La séance est reprise. Mes chers collègues, en raison de l'hommage national en mémoire des militaires français morts au Mali, qui se tiendra lundi 2 décembre après-midi aux Invalides, nous pourrions ne reprendre nos travaux l'après-midi qu'à dix-huit heures. Y a-t-il des observations ? Il en est ainsi décidé. En conséquence, en accord avec le Gouvernement, la commission des finances et les commissions concernées, l'examen de la mission « Travail et emploi », initialement inscrite le lundi 2 décembre, serait reporté au vendredi 6 décembre, en premier point de l'ordre du jour du matin.

Les délais limites pour les inscriptions de parole, ainsi que pour les cosignatures d'amendements, seraient quant à eux reportés au jeudi 5 décembre, à onze heures. Y a-t-il des observations ?

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, cette année encore est marquée par d'importants dérapages en matière de maintien de l'ordre ; et ces derniers montrent, une fois de plus, l'importance de la mission « Sécurités

L'année 2019 est également marquée par l'émergence d'un malaise particulièrement fort. Ce dernier s'est exprimé au cours de la grève intersyndicale du 2 octobre dernier, dont l'ampleur s'est révélée c'est la première fois depuis vingt ans que toutes les organisations syndicales ont manifesté ensemble. C'est dans ce contexte que nous abordons l'examen du budget 2020, qui n'est pas à la hauteur des enjeux.

Si l'on tenait compte de la réalité des modifications de périmètre, la hausse des crédits serait même plus soutenue : elle s'élèverait à 4,22 % en autorisations d'engagement et à 5,35 % en crédits de paiement pour le programme « Police nationale à 3,51 % en autorisations d'engagement et à 2,35 % en crédits de paiement pour le programme « Gendarmerie nationale ». Pour autant, depuis plusieurs années maintenant, je dénonce l'augmentation constante de la part des dépenses de personnel dans l'ensemble des dépenses des deux forces. Ce budget connaît les mêmes travers que ceux des années précédentes, et ce de manière particulièrement aggravée : la la part des dépenses de personnel dans le total des dépenses va dépasser 90 % pour la police nationale et 85 % pour la gendarmerie nationale. Je vous rappelle qu'il y a quatorze ans la part des dépenses de personnel dans le total des crédits était encore inférieure à 80 %. Cette évolution ne me semble ni soutenable ni maîtrisée. procède à mon sens d'une vision purement politique, visant à mener les recrutements annoncés coûte que coûte, au détriment de la capacité opérationnelle des forces, laquelle ne peut être restaurée sans dépenses de fonctionnement et d'investissement dignes

de près de 9 %. Ce budget traduit donc une hausse importante des dépenses de personnel, en augmentation de 3,6 % pour la police nationale et de 2,5 % pour la gendarmerie nationale. Cette hausse s'explique principalement par le fort niveau des recrutements par l'ampleur des mesures indemnitaires. Une augmentation de 1 398 emplois à périmètre constant est prévue pour la police nationale en 2020,

Ces augmentations sont conformes aux annonces présidentielles du début de quinquennat. Le coût de ces recrutements, pour 2019 et 2020, devrait s'élever dans le prochain budget à 47,45 millions d'euros pour la police nationale et à 16,36 millions d'euros pour la gendarmerie nationale. L'année 2020 devrait également être marquée par le poids budgétaire des mesures catégorielles prises en faveur des policiers et des gendarmes, en particulier avec la prime « gilets jaunes » du 27 décembre 2019. Ces dernières s'élèveront à 192 millions d'euros pour les premiers et à 91 millions d'euros pour les seconds. De manière parfaitement prévisible, et, comme ce fut le cas l'an dernier, la mission « Sécurités » dépassera de nouveau largement la trajectoire fixée par la loi de programmation des finances publiques : elle l'excédera d'environ 500 millions d'euros, ce qui représente près de 4 % des crédits de paiement exprimés en norme pilotable. norme pilotable. Elle fait ainsi partie des six missions présentant le plus fort dépassement par rapport à la loi de programmation des finances publiques. Ce dépassement résulte presque intégralement de l'absence de maîtrise des dépenses liées au personnel. Les dépenses d'investissement et de fonctionnement ont, quant à elles, atteint un niveau plancher. Cette situation traduit l'absence totale de marge de manoeuvre résultant du dérapage des dépenses de personnel que je viens d'exposer. Pour la gendarmerie nationale, à périmètre constant, les dépenses d'investissement et de fonctionnement seront pour ainsi dire stables en crédits de paiement et connaîtront une hausse de plus de 6 % en autorisations d'engagement. Pour la police nationale, les dépenses de fonctionnement et d'investissement reculent de 8,8 % en autorisations d'engagement et de 0,8 % en crédits de paiement par rapport à l'an dernier. Les crédits affectés au renouvellement des véhicules, qui constituent à mes yeux un bon indicateur de la volonté de restaurer la capacité opérationnelle des forces de l'ordre, paraissent très insuffisants

constituent l'un des principaux outils des agents, notamment dans la gendarmerie nationale. Le budget d'acquisition de véhicules des deux forces représente seulement le tiers des mesures de revalorisation salariale octroyées aux forces de l'ordre en 2020. Avant de conclure, je tiens à mentionner quelques évolutions importantes en matière d'organisation. Des efforts notables de rationalisation sont entrepris, avec la création d'une direction du numérique et d'un service d'achat unifiés au sein du ministère.

L'année 2019 est également marquée par l'abandon de la vacation forte. Comme je l'annonçais depuis 2016, ce renoncement était inévitable. Il est donc regrettable que les difficultés liées à ce nouveau cycle de travail aient fait perdre trois années à l'institution policière, suscitant des espoirs et faisant naître des crispations entre les unités bénéficiant de ce cycle et les autres. Cette perte de temps est d'autant plus déplorable que, du fait de son caractère insoutenable,

il n'y a jamais eu aussi peu de décès sur les routes de France. On a dénombré 3 488 morts en France, départements et collectivités d'outre-mer compris, soit 196 de moins qu'en 2017. Suivant la même trajectoire baissière, l'accidentalité a enregistré une diminution de 3 %. Réjouissons-nous, à travers ces bons chiffres, de toutes les vies sauvées sur nos routes.

cette stabilité est difficile à apprécier compte tenu à la fois de la mise en place des 80 kilomètres à l'heure au milieu de l'année 2018 et des détériorations de radars entre l'automne 2018 et la mi-2019.

Enfin, à l'échelle de notre continent, la France se situe seulement dans la moyenne des pays de l'Union européenne et plusieurs de nos voisins, comme l'Allemagne ou encore le Royaume-Uni, affichent de meilleurs résultats : la France dispose donc encore d'une marge de progression.

C'est ce que permettra le nouvel indicateur créé à cet effet et intitulé « nombre de tués hors agglomération et hors autoroutes ».

dont les coûts d'organisation représentent plus de la moitié des crédits. La réforme de cet examen, lancée en 2014, devrait connaître un second souffle grâce aux dix mesures annoncées le 2 mai 2019 par le Premier ministre, dont l'objectif est de rendre le permis à point moins cher et plus accessible. Deux mesures, l'extension de la formation sur simulateur et la conversion facilitée du permis sur boîte automatique, sont déjà entrées en vigueur en juillet 2019. Les autres le seront après la promulgation de la loi d'orientation sur les mobilités. Par ailleurs, alors que les indicateurs de performance stagnaient, le PLF 2020 a remplacé le délai moyen d'attente par le délai médian, qui devrait mieux refléter la baisse des délais pour la majorité des candidats.

Il s'agit là, à mon sens, d'une estimation optimiste : le montant du produit qui sera réalisé en 2019 est estimé à 1,700 milliard d'euros

Cela tient notamment au fait que, comme vous le savez, de nombreux radars ont été vandalisés ou neutralisés. Plus de 10 000 dégradations ont ainsi été constatées en 2018 et 7 500 au 1 septembre 2019 ; le taux moyen de disponibilité des radars est passé de 93 % en 2017 à 88 % en 2018, pour s'établir à seulement 75 % en 2019. Dans ces conditions, l'impact sur les recettes de l'État a été immédiat et s'est répercuté sur les amendes radars, dont le produit sera, en 2020, encore inférieur à son niveau de 2017. L'objectif de déploiement a, certes, été revu à la baisse, alors qu'il avait déjà pris du retard au cours des années précédentes, passant de 4 700 à 4 400 équipements d'ici à la fin 2020, mais il comptera, en revanche, des équipements plus modernes, et notamment environ 1 200 radars tourelles, contre 400 qui devraient avoir été installés à la fin de 2019, permettant un contrôle plus étendu et moins prévisible. Sur ce point, le délégué à la sécurité routière nous a confirmé, lors de son audition, la capacité technique des entreprises sous-traitantes à installer 800 nouveaux radars tourelles au cours de l'année 2020. S'agissant des collectivités locales, je constate que les crédits du programme 754 augmentent sensiblement, d'environ 29 %, en 2020, malgré l'entrée en vigueur de la décentralisation du stationnement payant, qui avait justifié, l'an dernier, leur diminution. Cette hausse s'explique par le dynamisme des amendes forfaitaires majorées et hors radars. Enfin, j'achèverai mon propos en évoquant sur la complexité de ce compte d'affectation spécial. Alors que les recettes estimées pour 2020 sont supérieures à la réalisation de 2019, avec 1,837 milliard d'euros contre 1,7 milliard d'euros, cette augmentation profiterait en premier lieu au programme de désendettement de l'État, qui s'établit, pour 2020, à près de 32

situation est totalement aberrante, dans la mesure où cette agence a pour mission le financement de programmes d'investissement ferroviaires, routiers et fluviaux, qui nécessitent une programmation stabilisée dans la durée. Le manque de lisibilité et de cohérence de ce système est devenu tellement contre-productif que l'État a présenté, dans le projet de loi de finances rectificative pour 2019, un article visant à réaffecter une partie du flux en provenance des amendes forfaitaires radars, initialement destiné à l'État et aux collectivités, vers le budget de l'Afitf.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le présent projet de loi de finances prévoit une diminution des crédits du programme 161, « Sécurité civile », par rapport à 2019, avec 519,5 millions d'euros de crédits de paiement prévus en 2020. Cette diminution s'explique essentiellement par une réduction du périmètre du programme 161, avec le transfert d'environ 15 millions d'euros de ses crédits vers le programme 216, « Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

Leurs dépenses d'investissement ont même connu une baisse importante, de près de 18 % depuis dix ans, qui est d'autant plus préoccupante que le soutien de l'État s'amoindrit d'année en année : la dotation de soutien aux investissements structurants des SDIS ne représente plus que 7 millions d'euros en 2020, contre 25 millions d'euros en 2017. De plus, cette dotation n'accordera plus aucun crédit en faveur des projets locaux des SDIS en 2020. J'estime qu'un effort financier de l'État aurait été possible, alors que les crédits du programme 161, notamment ses dépenses d'intervention, sont inférieurs de 10 millions d'euros à la programmation. J'achève mon propos par un dernier motif de préoccupation : plus d'un an et demi s'est écoulé depuis l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne. Ma collègue Catherine Troendlé et moi-même vous avions exhorté, monsieur le ministre, à en tirer les conséquences, car nous nous redoutons tous la menace qu'il fait peser sur notre système de volontariat des sapeurs-pompiers. Un an plus tard, il est regrettable que nous soyons toujours dans l'attente d'une initiative claire de la part du Gouvernement, alors que plusieurs recours ont été déposés devant les tribunaux administratifs. Une action rapide doit être entreprise, monsieur le ministre : allez-vous soutenir le projet d'une nouvelle directive qui semble, à nos yeux, la seule solution pour garantir la pérennité de notre modèle de sécurité civile ? ? J'ajoute quelques remarques à la suite de mon rapport sur la lutte contre les feux de forêt. Il est satisfaisant que ce projet de loi de finances prévoie toujours le remplacement des Tracker vieillissants par de nouveaux Dash. La livraison de ces avions me paraît toutefois tardive. Nous ne pouvons pas tolérer une éventuelle rupture capacitaire ces prochaines années, alors que le risque de feux de forêt est susceptible de s'aggraver. Deux de mes recommandations visaient donc à accélérer la livraison de ces Dash et à faire aboutir au plus vite les négociations européennes en vue d'une commande mutualisée de Canadairs. Je ne puis que réitérer ces recommandations devant vous, monsieur le ministre, indépendamment des incidents techniques qui peuvent immobiliser nos appareils pendant plusieurs mois. Vous me voyez d'ailleurs satisfait que nos sept Tracker soient de nouveau autorisés à voler depuis la semaine dernière. Leur participation aux missions de guet aérien armé reste essentielle, dans l'attente de leur remplacement par des Dash. Pour finir, je dois vous avouer ma déception concernant l'évolution du service d'alerte et d'information des populations, Ce projet de loi de finances pour 2020 marque le début de la seconde période de financement, qui représentait initialement 36,8 millions d'euros pour la période 2020-2022. Cette enveloppe a été réduite à 5,6 millions d'euros, qui financeront exclusivement la rénovation des sirènes. comment justifiez-vous une telle obstination en faveur de ce procédé, au détriment du développement d'un système d'alerte par téléphone ? Un tel système était pourtant préconisé dès le Livre blanc de 2008 et devient, plus que jamais, indispensable dans un pays comme le nôtre. Les récents exemples de l'incendie de l'usine de Lubrizol et des intempéries dans le Sud-Est en ont fait la démonstration : une technologie de diffusion cellulaire, le, aurait été bien plus efficace et aurait permis une alerte claire et immédiate. En outre, une directive européenne nous impose la mise en place d'une transmission des alertes par téléphone d'ici à 2022. Vos services, monsieur le ministre, affirment que cette obligation est en cours de réalisation. Comment se fait-il, alors, qu'aucun crédit, ni en CP ni en AE, ne soit prévu pour le développement d'un quelconque volet mobile, ni dans ce PLF, ni pour 2021, ni pour 2022 ? Pour conclure, mes chers collègues, l'ensemble de ces préoccupations m'incite à vous proposer le rejet de ces crédits.

Connaissez-vous, monsieur le ministre, le « Bon Coin des gendarmes » ? C'est une sorte de bourse où ces derniers s'échangent des pièces de rechange ou des objets qui leur permettent, tout simplement, de continuer à remplir leurs missions malgré la pénurie de moyens

Quant aux crédits prévus pour les réservistes, qui sont désormais essentiels au plein accomplissement des missions de la gendarmerie, ils seront également, une fois de plus, en forte baisse en 2020. La gravité de la situation s'explique non seulement par une insuffisance des crédits, mais aussi, plus que jamais, par la réserve de précaution, ce mécanisme, auquel s'ajoute le surgel ministériel, est en effet particulièrement dommageable pour la gendarmerie, dont une grande part des dépenses sont contraintes, comme le paiement des loyers ou des fluides. Ce sont donc les véhicules et l'immobilier, dont les crédits sont déjà calculés au plus juste, qui sont affectés massivement par ce gel. Avez-vous des pistes, monsieur le ministre, pour résoudre cette difficulté majeure que le directeur général de la gendarmerie évoque chaque année ? dernier sujet que je souhaite aborder est celui de la présence territoriale de la gendarmerie. Certaines propositions formulées à l'issue des ateliers d'idéation du début de l'année peuvent inquiéter, d'autant que nous savons qu'elles sont qu'elles sont tout à fait prises au sérieux. J'ai en particulier à l'esprit la réduction de plus du tiers du nombre de brigades, au moment où les Français réclament avec force plus de services publics dans nos territoires.

de sécurité, des moyens et une organisation en accord avec leur mission, la commission a émis un avis défavorable à l'adoption des crédits du programme « Gendarmerie nationale ». La parole

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je voudrais commencer par rendre hommage à nos gendarmes, qui ont dû faire face à des situations particulièrement difficiles en 2019, en matière de maintien de l'ordre, notamment face à quelques éléments du mouvement des « gilets jaunes ». Je reviens sur les propos de Philippe Paul, qui a évoqué l'éventualité d'une loi de programmation. Nous savons que des travaux d'élaboration d'un Livre blanc de la sécurité intérieure sont en cours. Or il est essentiel que ce Livre blanc se traduise, ensuite, par une loi d'orientation et de programmation. Nous l'avons fait pour la défense, nous devons le faire pour la sécurité intérieure Il est indispensable que cette future loi comporte une programmation financière mettant en adéquation les moyens de la gendarmerie et de la police nationale avec leurs missions. Monsieur le ministre, est-ce bien ce qui est prévu ? prévu ? Il existe actuellement un écart de plus en plus douloureux entre ce qui est demandé à nos gendarmes et les outils qui sont mis à leur disposition. S'agissant des véhicules,

malheureusement identique : avec une baisse des crédits en 2020, nous sommes très loin des 300 millions d'euros devant être dégagés annuellement pour entretenir décemment le parc domanial. Les gendarmes sont particulièrement affectés par cette insuffisance qui touche, bien sûr, leurs familles.

Mes chers collègues, nous en sommes tous conscients, nos forces de sécurité ont besoin d'être fortement soutenues dans une période difficile, dans laquelle, après avoir été encensées à la suite des attentats, elles sont parfois la cible de mécontentements diffus. Ainsi, au 30 juin de cette année, la gendarmerie a enregistré une augmentation de 11,5 % des agressions physiques par rapport à l'an passé, une hausse de 3,7 % du nombre de blessés à la suite d'agressions armées et une progression de 11,4 % du nombre de blessés à la suite d'agressions sans arme. Parce que nous soutenons nos gendarmes, il est indispensable que, avec l'accroissement des effectifs, soit entreprise une augmentation plus importante des crédits consacrés au matériel, ainsi qu'une amélioration globale de leurs conditions de logement. Merci par avance, monsieur le ministre, de les entendre, après nous avoir écoutés

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, depuis plusieurs exercices, notre commission regrette, en dépit des efforts consentis pour le budget de la sécurité, l'approche déséquilibrée du Gouvernement, qui privilégie le renforcement des effectifs au détriment de l'amélioration des conditions de travail des policiers et des gendarmes. Alors même que les revendications de nos forces de l'ordre n'ont jamais été aussi fortes, le projet de loi de finances pour 2020 ne déroge malheureusement pas à la règle. à la règle. Pour aller à l'essentiel, j'insisterai sur trois sujets d'inquiétudes soulevés par notre commission. Le premier concerne les crédits d'investissement, qui chuteront, à périmètre constant, de 13,6 % dans la police et de 17,4 % dans la gendarmerie. Cette année encore, monsieur le ministre, le compte n'y est pas : comment espérez-vous garantir à nos forces une modernisation de leurs parcs automobiles et améliorer leur situation immobilière avec des dotations en baisse ? J'ai déjà eu l'occasion de le dire dans cet hémicycle il est illusoire de penser qu'augmenter le nombre de nos policiers et de nos gendarmes suffira à renforcer leur capacité opérationnelle, si l'on n'entretient pas, dans le même temps, leurs moyens d'intervention. Le deuxième sujet concerne le financement des réserves de la police et de la gendarmerie. Depuis deux ans, les enveloppes qui leur sont allouées sont systématiquement ponctionnées, pour financer les recrutements et les mesures de revalorisation salariale.

Ces coupes budgétaires risquent d'appauvrir, à terme, le vivier des réservistes, dont l'appui aux forces de sécurité est pourtant devenu essentiel. Enfin, je dirai quelques mots sur les conséquences des nombreuses créations de postes souhaitées par le Gouvernement sur les dispositifs de recrutement et de formation de la police et de la gendarmerie. Pour absorber l'augmentation des entrées en école, les dispositifs de formation ont été adaptés, parfois dans l'urgence, avec des conséquences qu'il est encore difficile d'évaluer. Il est heureux que des mesures de plus long terme aient été prises pour renforcer durablement la capacité d'accueil des écoles, mais j'ai pu constater qu'il existait un risque réel de saturation. Au-delà de l'insuffisance des budgets de fonctionnement des écoles, c'est surtout l'appauvrissement des viviers de recrutement et la baisse des niveaux de sélectivité des concours qui inquiètent, à juste titre, nos collègues. Monsieur le ministre, il ne suffit pas de recruter en nombre ; il s'agit aussi de recruter en qualité. À défaut, c'est la sécurité des Français que vous risquez de dégrader encore plus. Vous l'avez compris, la commission des lois a émis, à la lumière de ces éléments, un avis défavorable à l'adoption des crédits de la mission « Sécurités » hors programme « Sécurité civile ». La

ne disposant que de trois minutes, je ne vais pas décrire ce budget qui stagne ou répéter que la sécurité civile est devenue le parent pauvre de la sécurité. Nous le savons tous. Je vais aller à l'essentiel en évoquant deux points, à commencer par les suites de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne. Cette décision a reconnu la qualité de travailleur à un sapeur-pompier volontaire belge et pourrait remettre entièrement en cause notre modèle de sécurité civile. Lors de son audition, Laurent Nunez a indiqué vouloir exploiter les dérogations offertes par la directive de 2003 sur le temps de travail pour nous sortir de l'ornière.

pérenne est l'adoption d'une directive européenne, destinée à l'engagement citoyen. Un projet est déjà rédigé ; il n'attend que votre soutien, monsieur le ministre. Mon deuxième point concerne l'investissement des SDIS. En 2016, la réforme de la prestation de fidélisation et de reconnaissance (PFR) versée aux sapeurs-pompiers volontaires s'est traduite par une diminution significative du montant de la participation versée à ce titre par l'État aux départements, en contrepartie de l'abondement d'un fonds à hauteur de cette économie, dédié au soutien aux investissements structurants des SDIS. L'idée était de rendre à la sécurité civile ce qui lui appartenait déjà. Cet engagement logique n'a tenu qu'une seule année : depuis lors, les économies restent, mais le montant du fonds n'a, quant à lui, cessé de diminuer. Sur quatre ans, la différence s'élève à 60 millions d'euros, soit plus de 10 % du budget annuel de la sécurité civile. Comment expliquer cette baisse, alors que les investissements des SDIS sont au plus mal et que le budget du programme « Sécurité civile » ne représente que 2,5 % de celui de la mission « Sécurités

monsieur le ministre, vous annonciez un plan en faveur de la sécurité des sapeurs-pompiers. La commission des lois du Sénat s'intéresse également à ce sujet central et la mission d'information qu'elle a créée, dont je suis corapporteur, rendra son rapport le 11 décembre. Monsieur le ministre, la sécurité de nos sapeurs-pompiers est largement tributaire de la qualité des équipements qui les protègent. Aussi, mes collègues corapporteurs et moi-même vous demandons un geste simple, évident, frappé au coin du bon sens : rendez à la sécurité civile et aux pompiers l'argent qu'ils vous ont fait économiser et fléchez cette somme, en priorité, vers les investissements nécessaires pour assurer leur sécurité. Je vous laisse compter combien de parebrises feuilletés, de caméras piétons et de gilets pare-lames on achète avec 60 millions d'euros

pas réglé. Mes chers collègues, je vous rappelle que le temps de parole attribué à chaque groupe pour chaque unité de discussion comprend le temps de l'intervention générale et celui de l'explication de vote.

Monsieur le ministre, nous sommes à votre écoute pour savoir comment vous entendez poursuivre l'opération de résorption des heures supplémentaires et gérer les récupérations et les prises de congés de manière que l'ambiance sociale,

pas là où nous l'attendions. S'agissant du budget des forces de sécurité, le Gouvernement s'entête dans un choix qui a pourtant fait les preuves de son inefficience, renforçant les effectifs de police et de gendarmerie, d'un côté, avec la création de 1 888 emplois supplémentaires, tout en négligeant, de l'autre, leurs conditions de travail, avec des dotations de fonctionnement et d'investissement sous-budgétées. Certes, le recrutement au sein de la police nationale et de la gendarmerie ne cesse d'augmenter, d'augmenter, mais à quel prix et dans quel but ? À lire les observations du rapporteur spécial de la commission des finances, je ne suis guère rassurée : « l'évolution des dépenses de personnel des programmes " Police nationale " et " Gendarmerie nationale " n'apparaît ni soutenable ni maîtrisée ». La commande purement politique de ces schémas d'emplois apparaît même largement contre-productive et en totale inadéquation avec les besoins de nos forces de l'ordre, puisque, si les dépenses de fonctionnement et d'investissement sont en diminution, atteignant un niveau plancher, cela résulte toujours, selon le rapporteur spécial, « du dérapage des dépenses de personnel ». Pour compenser la hausse des effectifs et les mesures d'accompagnement des policiers en 2020, monsieur le ministre de l'intérieur, vous taillez donc dans les dépenses d'équipement et d'investissement des forces de l'ordre, alors même que la hausse des dépenses de personnel du ministère de l'intérieur avait déjà été sévèrement taclée par la Cour des comptes dans son rapport sur l'exécution du budget de 2018. Les magistrats mettaient même en garde contre un effet de ciseau obligeant la place Beauvau à sabrer dans les budgets d'équipements, au risque d'affecter la capacité opérationnelle des troupes.

mais bien pour une amélioration de leurs conditions de travail et la défense de leurs retraites, ainsi que pour une loi de programmation ambitieuse pour un service public de qualité. Or les dépenses de fonctionnement en autorisations d'engagement diminuent de 16 %, quand les dépenses d'investissement chutent de 23 %.

une première réponse, très attendue, à la souffrance des pompiers, confrontés à un écart grandissant entre l'accroissement des missions et la stagnation des effectifs.

Monsieur le président, monsieur le ministre, madame, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues,

réels, ces efforts paraissent bien modestes au regard du contexte sécuritaire, particulièrement tendu, et n'apportent pas de réponse satisfaisante à la dégradation des conditions de travail des policiers et des gendarmes. En effet, la prégnance de la menace terroriste, l'importance de la pression migratoire à laquelle notre pays fait face depuis, désormais, plus de quatre ans et le maintien d'un niveau élevé de délinquance impliquent une mobilisation sans précédent des forces de sécurité intérieure sur notre territoire. Si les effectifs des forces de police et de gendarmerie ont été renforcés au cours des derniers exercices budgétaires, des efforts restent à fournir en ce qui concerne les moyens matériels pour parvenir au niveau exigé par l'aggravation de la situation. L'effort budgétaire demeure toujours en deçà des attentes et des besoins des forces de sécurité intérieure, dont les conditions matérielles continuent de se dégrader. La hausse des crédits paraît très insuffisante aussi compte tenu des violences urbaines récurrentes auxquelles les forces de l'ordre sont aujourd'hui confrontées.

au vieillissement des parcs automobiles de la police et de la gendarmerie ni de poursuivre la remise à niveau des équipements des forces de sécurité. Il ne permettra pas non plus la rénovation du parc immobilier, souvent dans un état de délabrement avancé. L'importante dégradation de la situation matérielle de nos forces de sécurité contribue bien évidemment au mal-être croissant au sein de la police et de la gendarmerie nationales.

la priorité donnée aux dépenses de masse salariale pèse fortement sur les dotations de fonctionnement et d'investissement, qui continuent globalement à diminuer. Avant de conclure, je souhaite rendre hommage, à cette tribune, aux hommes et aux femmes qui, tous les jours, souvent au péril de leur vie, veillent sur notre sécurité. Je salue leur engagement au service de nos concitoyens. Monsieur le ministre, votre budget ne prévoit pas suffisamment de moyens matériels pour la police et la gendarmerie nationales. Il ne prend pas assez la mesure de la dégradation du contexte sécuritaire dans notre pays. Même si des actions sont menées

plus de 20 000 personnes ont été suivies et 2 594 prises en compte. Quant aux salles de prières radicales salafistes,

nationale : la police de sécurité du quotidien et la sécurisation d'événements heureux, comme l'organisation de la coupe du monde de rugby en 2023. Depuis le début du quinquennat, conformément à l'engagement présidentiel, les lois de finances successives ont renforcé la situation financière du ministère de l'intérieur au regard de l'ensemble du budget de l'État. À ce rythme, la promesse de 10 000 renforts supplémentaires devrait être tenue, même si des effets de bords sont difficiles à anticiper, parce qu'ils dépendent de choix individuels- je pense en particulier aux demandes de départ anticipé à la retraite. Le Gouvernement propose une double réponse à la question des heures supplémentaires,

Il est bon que, enfin, l'État règle ses dettes auprès de ceux qui le servent ! L'effort du Gouvernement en ce sens est indéniable et remarquable au regard des exercices pré-attentats. Il est vrai que cet effort budgétaire accompagne une mobilisation exceptionnelle de nos forces de l'ordre, après leur engagement sans faille à la suite des attentats de 2015. Personne ne contestera en outre que, depuis un an à présent, l'encadrement du mouvement hebdomadaire des « gilets jaunes » s'est traduit par un investissement humain supplémentaire et a nécessité l'adaptation des techniques de maintien de l'ordre pour permettre à des fonctionnaires de police non formés à l'exercice de s'y intégrer. L'intensité de ces urgences récurrentes est mal vécue sur le terrain et déborde sur la vie familiale des agents mobilisés. Une désescalade doit intervenir ; au reste, elle commence déjà à se faire sentir. Elle passera notamment par un retour à la normale en termes de dialogue social, par l'intermédiaire des syndicats, mais aussi par des modalités de manifestation plus classiques, comme la mobilisation annoncée pour le 5 décembre prochain. Pour le reste, le Parlement a récemment adopté une loi renforçant considérablement les moyens de lutte contre les Black Blocks, qui devrait également produire des effets. Au regard de ces éléments et de l'évolution des indices de l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales, le budget proposé pour la mission « Sécurités » nous paraît crédible. Bien sûr, on peut toujours arguer que l'on pourrait faire mieux, avec plus de moyens ... Mais, comme l'a souligné Henri Leroy, rapporteur pour avis, l'accélération des recrutements de forces de l'ordre comporte également un risque de recrutement de moindre qualité, qu'il ne faudrait pas prendre à la légère. nous sommes très attachés à ce que l'ordre républicain soit incarné par des fonctionnaires. C'est pourquoi nous considérons avec scepticisme les évolutions vers un continuum de sécurité qui s'étendrait aux forces de sécurité privées, évolutions proposées par certains de nos collègues députés.

Sur le plan humain toujours, la politique de mobilité des agents du ministère de l'intérieur devrait faire l'objet d'une réflexion particulière, s'agissant de professions particulièrement usantes. Je n'oublie pas que, depuis le début de l'année, plus de cinquante agents se sont donné la mort. Nous espérons que ces préoccupations trouveront des réponses dans la loi de programmation qui a été annoncée, et que celle-ci permettra d'adapter définitivement l'organisation du temps de travail aux normes européennes. Nous serons d'ailleurs vigilants quant aux conséquences budgétaires de la réduction infligée à la sécurité civile. Par ailleurs, nous nous satisfaisons que les moyens alloués à la sécurité routière soient préservés, comme notre excellent collègue Jean-Marc Gabouty l'a souligné. Nous estimons en effet que la sécurité routière doit passer par l'éducation et l'amélioration des équipements routiers,

Pourquoi s'entêter à installer nos administrations dans la région la plus chère de France ? Dans le même esprit, il peut paraître paradoxal d'équiper nos gendarmes de terminaux ultrasophistiqués qu'ils auront sûrement de la peine à utiliser dans les zones blanches de notre territoire ... Le droit à la sécurité doit être assuré partout ! Malgré ces quelques observations, notre groupe ne s'opposera pas à l'adoption des crédits de la mission

Les grandes métropoles frontalières connaissent des problèmes de sécurité, et les élus locaux sont en première ligne pour recevoir et entendre les doléances des habitants. Répondons-nous vraiment à leurs attentes, à leurs constatations jugées prioritaires Une augmentation progressive des trafics de stupéfiants est observée depuis des années, qu'il s'agisse de leur ampleur, du nombre de sites touchés ou de la diversité des substances écoulées. Plusieurs kilogrammes de cocaïne ont été trouvés échoués sur les plages françaises : c'est invraisemblable Les trafics sont le principal fléau des quartiers, et les habitants en sont les premières victimes, subissant les nuisances, les dégradations, les squats et, souvent, les violences de ceux qui tiennent les marchés des stups.

ministre, le nombre de policiers a été renforcé, et, je vous l'accorde, vous avez décidé de faire face à cette délinquance massive qui pollue l'évolution des banlieues et anéantit l'avenir des enfants des cités. Certes, les préfets sont réactifs, organisant, en liaison avec les élus locaux, des lieux de concertation pour cerner les problèmes de sécurité. Certes, l'éducation nationale, les services socioéducatifs, les bailleurs sociaux et toutes les institutions concernées par l'insécurité mettent en place de vraies politiques pour les zones de sécurité prioritaire. Reste à gérer le problème de l'organisation des ressources humaines. Tant de policiers et de gendarmes sont accaparés, chaque semaine, par la tension sociale. Combien d'hommes et de femmes sont depuis un an au coeur des manifestations à maintenir l'ordre, policiers et gendarmes qui ne sont plus disponibles sur le terrain pour enrayer la petite et moyenne délinquance ? Que dire aussi de la situation dans les prisons, où les gardiens, débordés et manquant de moyens, doivent faire face à une violence toujours plus exacerbée ?

Un colonel de sapeurs-pompiers nous disait, lors d'une réunion de sécurité, que, même en situation de guerre, on respectait jusqu'alors l'intégrité des ambulances ... Aujourd'hui, Les pompiers, héros du quotidien, ne peuvent pas être abandonnés sur le terrain, alors qu'ils mettent leur vie en jeu pour sauver celles des autres. Monsieur le ministre, Aujourd'hui, nous attendons que le budget « Sécurités » soit à la hauteur de l'évolution de la violence. Augmenter le nombre de policiers n'est pas une fin en soi, surtout

sécurité. La création de près de 2 000 emplois supplémentaires dans la police et la gendarmerie n'a pas de sens, si ces recrutements sont opérés au détriment de l'équipement.

Les locaux dans lesquels travaillent nos fonctionnaires de police sont trop souvent vétustes et parfois même dangereux du point de vue sanitaire, pour les policiers comme les justiciables. Par ailleurs, les réserves de la police et de la gendarmerie, qui assurent un lien entre les citoyens et leurs forces de sécurité, sont elles aussi victimes de coupes budgétaires importantes. Monsieur le ministre, il est grand temps d'apporter à tous ceux qui assurent la sécurité de nos concitoyens une réponse globale aux problèmes auxquels ils font face. Malheureusement, votre budget n'est pas à la hauteur,

très difficile. L'une des principales sources de l'insécurité est le terrorisme. À cet égard, monsieur le ministre, nous avons tous en mémoire le drame qui s'est produit à la préfecture de police de Paris

les crédits alloués à l'action Commandement, ressources humaines et logistique baissent de 16,87 % en autorisations d'engagement

Plus de 1 000 policiers et plus de 490 gendarmes renforceront l'année prochaine les capacités de notre pays. Ce n'est pas rien. Au moment où notre pays poursuit aussi son effort de remontée en puissance un exécutant la loi de programmation militaire, le cap du régalien est tenu, qu'il s'agisse du respect de l'ordre public ou de la souveraineté de la France. Pour la police, la progression est plus marquée pour l'action n° 01, Ordre public et protection de la souveraineté, et l'action n° 04, Police des étrangers et sûreté des transports internationaux. Cette progression

La commission des lois a estimé que la montée en puissance des dépenses de fonctionnement limitait à l'excès les crédits alloués à l'équipement des forces de sécurité ; le

pris en matière de revalorisation des carrières, d'amélioration des rythmes de travail et, plus généralement, de charges de service,

avec laquelle il les met en oeuvre ... J'espère que les nouveaux moyens ouverts en matière de sécurité permettront d'améliorer les conditions de recrutement, sujet sur lequel

Monsieur le président, monsieur le ministre, madame, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, le général L'Hotte, écuyer en chef du Cadre noir, répondait chaque matin, à qui lui demandait comment il allait : « Calme, en avant et droit ». C'est dans cet état d'esprit que j'aborderai le sujet majeur de la mission « Sécurités » dans le cadre du PLF 2020. Mes chers collègues, rendons hommage à nos forces de l'ordre. Il m'apparaît essentiel de rappeler que nos forces de sécurité civiles et militaires ont vécu une année 2019 extrêmement éprouvante, avec une mobilisation sur tous les fronts : « gilets jaunes », prévention face à la menace terroriste, sécurité des biens et des personnes, impact psychologique face à la nouvelle violence de la rue et haine « anti-flic ». Manque d'effectifs, commissariats et casernes vétustes, véhicules obsolètes : les gendarmes et les policiers réclament un plan Marshall de la sécurité intérieure. Le nombre important de suicides, tant dans la police que dans la gendarmerie, témoigne malheureusement de l'état psychologique dégradé de nos forces de sécurité, qu'il est urgent de protéger. Les quatre programmes de la mission- « Police nationale », « Gendarmerie nationale », « Sécurité civile » et « Sécurité et éducation routières » -soutiennent les actions spécifiques et conjointes des acteurs de la sécurité intérieure.

Comme lors de l'examen des précédents projets de loi de finances, l'approche du Gouvernement privilégie le renforcement des effectifs au détriment de l'entretien des équipements et des moyens d'intervention. Mais quel est le bon choix ?

Sachant que l'efficacité des policiers et gendarmes repose non pas uniquement sur leur nombre, mais également sur la qualité de leur équipement, on peut en déduire que l'augmentation continue des effectifs, sans augmentation des dépenses de fonctionnement et d'investissement, risque de nuire à leur capacité opérationnelle. C'est tout le indique que l'engagement de la gendarmerie et de la police restera guidé par la lutte contre toutes les formes de délinquance, la présence sur le terrain et la proximité avec la population, ce qui est fondamental. Dans le cadre de la police de sécurité du quotidien, la gendarmerie et la police devraient poursuivre la mise en oeuvre de stratégies locales sur des territoires à forts enjeux de sécurité. En ce qui concerne la sécurité civile, le rapporteur a considéré qu'elle était devenue la parente pauvre du budget de la mission : les crédits stagnent, les emplois baissent. Il n'y a aucune perspective d'évolution à moyen terme. Les investissements des SDIS sont toujours en souffrance et ne sont quasiment plus soutenus par l'État. Encore au stade de la préfiguration, la montée en puissance du service national universel, le SNU, qui associe les SDIS, fait craindre un nouveau transfert de charges de l'État vers les collectivités. En ce qui concerne la sécurité et l'éducation routières, le PLF met en avant le lien entre les bons résultats en termes de mortalité routière et l'abaissement de la vitesse maximale de 90 à 80 kilomètres Mais il peut être très difficile d'apprécier précisément les effets d'une telle mesure. Mon collègue, Jean Marc Gabouty, rapporteur spécial, atteste que l'année 2019 a représenté l'un des plus bas niveaux historiques de décès sur la route.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, mon intervention portera sur les crédits accordés à la sécurité civile au sein de la mission « Sécurités Pour l'année 2020, ces crédits sont en baisse de 3,3 % par rapport à la dotation de l'exercice précédent, voire de plus de 4 % en tenant compte des perspectives d'inflation pour 2019. Cette diminution s'explique par le transfert des crédits liés aux systèmes d'information et de communication vers le programme 216. Toutefois, même en neutralisant les effets de ce changement de périmètre, les crédits de paiement du programme 161 marquent le pas. C'est d'autant plus regrettable que le budget de la sécurité civile représente seulement 2,5 % des crédits dévolus à la mission « Sécurités ». Je souhaite également souligner que ce budget ne représente qu'une faible part des 6 milliards d'euros consacrés chaque année à la sécurité civile en France,

je tiens à mon tour à rappeler la menace que fait planer l'arrêt, rendu le 21 février 2018 par la Cour de justice de l'Union européenne, qui assimile les sapeurs-pompiers volontaires à des travailleurs et qui plafonne à 2 304 heures par an Ceux d'entre eux qui exercent une activité salariée principale à temps plein ne pourraient donc plus consacrer que 697 heures par an à leurs activités de sapeurs-pompiers volontaires. cet arrêt assimilant leurs périodes d'astreinte à du temps de travail, c'est la viabilité même de notre modèle français de sécurité civile qui est remise en cause. Mon département du Finistère compte ainsi 465 sapeurs-pompiers professionnels pour plus de 2 000 sapeurs-pompiers volontaires, qui ont choisi de s'engager en sus de leurs heures de travail et ont accepté, à cette fin, de suivre une formation exigeante et contraignante. Je souhaiterais Je souhaiterais donc savoir, monsieur le ministre, de quelle manière vous envisagez les discussions sur ce sujet avec la nouvelle Commission européenne. Il y a urgence ! Les SDIS doivent en outre faire face à un accroissement continu des sollicitations opérationnelles. Leur volume annuel d'interventions a ainsi augmenté de 25 % entre 2003 et 2017. Sur la même période, les incendies ne représentaient plus que 7 % de leur activité, tandis que les secours à la personne connaissaient une augmentation de 64 %. Les sapeurs-pompiers sont donc confrontés à une véritable mutation de leur métier. Ils sont notamment amenés à compenser les conséquences des restructurations sanitaires et de la diminution des permanences médicales de proximité. le secours d'urgence à la personne est devenu l'activité principale des SDIS, en particulier dans les territoires touchés par la désertification médicale. La Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France estime ainsi qu'ils assument, à eux seuls, près de 95 % des urgences pré-hospitalières. Par ailleurs, je tiens à déplorer la hausse des violences exercées à l'encontre des sapeurs-pompiers qui accentue encore un peu plus le malaise de cette institution d'après l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales, entre 2008 et 2017, le taux d'agressions déclarées a augmenté de 213 %. Sur ce sujet, je me félicite de ce que le Sénat ait adopté, en mars dernier, la proposition de loi de Patrick Kanner et du groupe socialiste et républicain visant à renforcer la sécurité des sapeurs-pompiers, même si ses dispositions ont été amoindries.

Il s'agit toutefois d'une première avancée indéniable. Ce texte a également permis la création, en avril 2019, d'une mission sénatoriale sur la sécurité des sapeurs-pompiers, dont les conclusions viendront enrichir notre action. En tout état de cause, l'État se doit, au préalable, de garantir des moyens à la hauteur des besoins de notre sécurité civile. Ce n'est pas le cas dans ce projet de budget : au-delà des chiffres que j'ai évoqués précédemment, la dotation de soutien aux investissements des SDIS passera de 25 millions d'euros en 2017 à seulement 7 millions pour 2020 ! Pis, aucun de ces crédits ne sera accordé en faveur des projets locaux des SDIS. Ce n'est pas acceptable.

Ce budget doit permettre de poursuivre le recrutement de 1 465 policiers supplémentaires en 2020 et d'améliorer leurs conditions de travail. Si nous avons privilégié les salaires, les crédits d'investissement et de fonctionnement ne sont pas en reste.

Les deux tiers de ces crédits seront consacrés à des dépenses de fonctionnement et d'investissement pour un montant de 347 millions d'euros. Les Trackers seront remplacés par des Dash neufs,

effet, si je prenais des décisions que d'autres paient, je pense que les sénateurs, défenseurs des collectivités, pourraient me le reprocher ... Je veux bien entendre le procès qui m'est fait, mais partons de ces réalités. Sur les chantiers qui relèvent du ministère de l'intérieur, comme celui des retraites, par exemple, nous avons travaillé avec les organisations syndicales. Les choses suivent leur cours et se passent bien,

une circulaire sur l'engagement qui irait bien au-delà de la question des sapeurs-pompiers, mais, vous le savez comme moi, il faudra l'accord de l'ensemble des pays européens, ce qui est un cheminement quelque peu compliqué.

à la sécurisation des plages des littoraux français. Cette participation est remise en cause, comme le souligne la Cour des comptes dans une communication de septembre 2012 devant la commission des finances de l'Assemblée nationale sur l'organisation du secours en montagne et de la surveillance des plages. Il s'agit d'un aspect peu connu

des vacanciers et des gens du pays que pour lutter contre la « délinquance du sable ». Dès 2012, la Cour des comptes constatait d'ailleurs l'indéniable progression des enjeux de sécurité publique, compte tenu d'une délinquance croissante sur les plages. Dans ce contexte sécuritaire plus sensible, il serait regrettable

dans les ressorts de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon de marins-pompiers de Marseille. Cette mesure me semble pertinente quant à l'objectif. Il s'agit Il s'agit en effet d'assurer sur l'ensemble du territoire la continuité de la prise en charge des victimes secourues par ces associations, jusqu'à leur transfert vers un établissement de santé. Cependant, le dispositif proposé n'a aucune incidence directe sur les charges de l'État et ne doit pas, dès lors, figurer dans la présente loi de finances, dont le domaine est encadré par l'article 34 de la loi organique relative aux lois de finances, la LOLF. Son adoption dans le texte définitif l'exposerait à une censure du Conseil constitutionnel. Par ailleurs, la rédaction de cet article soulève plusieurs difficultés et mérite d'être améliorée, afin de garantir notamment la pleine maîtrise des SDIS s'agissant du recours aux moyens complémentaires qu'offriraient ces associations dans leurs opérations de secours d'urgence aux personnes.

favoriser les politiques de prévention, conformément aux souhaits exprimés tant par le Gouvernement que par les usagers de la route et les associations de prévention de la sécurité routière. Il s'agit donc de transférer les crédits de l'action n° 01 du programme « Désendettement de l'État » vers l'action n° 01 du programme « Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières ».

On peut adhérer au souhait d'améliorer les équipements routiers des collectivités territoriales, mais le présent compte d'affectation spéciale doit, à mon avis, être totalement rebâti. Il serait sans doute souhaitable,

Je trouve que, dans une institution comme le Sénat, on ne devrait pas dire ça : les radars sauvent des vies ! S'il y a encore des femmes et des hommes pour penser que les limitations de vitesse n'ont pas sauvé de vies depuis que

Cet amendement vise à consacrer les recettes des « amendes radars » à l'amélioration du réseau routier et de ses zones les plus accidentogènes et, ainsi, à favoriser les politiques de prévention, conformément aux souhaits exprimés tant par le Gouvernement

programme « Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières ». Ces dépenses seraient ainsi limitées, d'une part, aux dépenses relatives à la conception, à l'acquisition, à l'entretien, à la maintenance et au développement des équipements des forces de sécurité

spécial. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, l'article 24 de la Constitution dispose que le Parlement vote la loi, contrôle l'action du Gouvernement et évalue les politiques publiques. En matière d'immigration, d'asile et d'intégration, il ne faut pas y compter : le Parlement doit voter à l'aveuglette, en se fondant sur des chiffres éparpillés dans de multiples missions, souvent artificiellement minorés ou majorés. Plutôt que de parler d'informations sans valeur, je voudrais donc profiter de ces quelques minutes pour quitter les chiffres et les détails techniques, et revenir aux principes. Le président Macron s'inquiétait récemment, dans, de « l'échec de notre modèle » d'intégration.

tout en condamnant à de la prison ferme les jeunes militants de Génération identitaire pour une fermeture symbolique des frontières françaises. Voilà qui est de nouveau faux ! Nous arrivons ici aux limites du « en même temps » cher au chef de l'État. À force de ne pas vouloir choisir, nous nous sommes enfoncés dans une impasse, et les risques de partition évoqués par François Hollande ou les risques de face-à-face violent envisagés par Gérard Collomb deviennent chaque jour plus vraisemblables. La première chose à faire, c'est évidemment de revenir à l'honnêteté et à la clarté. d'abord : il n'est pas admissible que la représentation nationale débatte dans un flou si peu artistique. Comme les années précédentes, les chiffres dont nous disposons pour cette mission sont notoirement biaisés.

: j'y ai découvert que la population de clandestins en Seine Saint-Denis variait, selon les estimations, de 150 000 à 400 000 personnes ! C'est au nom d'une conception angélique des droits de l'homme que nous nous interdisons toute connaissance précise des réalités démographiques et,, des coûts sociaux, économiques, culturels et politiques de l'immigration. Ce qui est certain, en tout cas, c'est que l'ensemble de ces coûts représente, comme dirait notre Président, un « pognon de dingue ». La clarté, ensuite. Nous avons besoin d'une politique migratoire claire et compréhensible par tous, Français comme étrangers. Comment comprendre que, en quelques mois, nous soyons passés du pacte de Marrakech et de son droit illimité pour tous à émigrer à un discours de fermeté, sans jamais remettre en cause ledit pacte ? Au-delà de la clarté et de l'honnêteté, deux vertus manquent cruellement pour que ce budget ait la moindre chance de répondre aux légitimes attentes de nos compatriotes : la cohérence et le courage. Je commencerai

surcroît, au moment même où la France devient le premier pays d'Europe pour les demandes d'asile, tant notre système est généreux avec l'argent de ces contribuables à qui nous demandons « en même temps » de se serrer la ceinture et d'accepter sans rien dire la préférence étrangère. Je fais partie, mes chers collègues, de ceux qui pensent, comme des hommes politiques aussi différents que Valéry Giscard d'Estaing, Georges Marchais ou Jacques Chirac, qu'il faut non seulement arrêter l'immigration illégale, bien sûr, mais aussi réduire drastiquement les plus de 400 000 entrées légales. Cependant, le plus impardonnable pour des responsables politiques, c'est le manque de courage. Il n'y a, en réalité, pas de politique migratoire en France, pas de volonté réelle de contrôler nos frontières ni d'intégrer les étrangers ou les Français récemment naturalisés sur notre sol. Allons-nous donc poursuivre notre absence de politique migratoire, refusant de regarder en face le tragique de l'histoire et oubliant délibérément ce qu'il en a coûté à nos aïeux de nous léguer un grand pays, libre et rayonnant sur le monde ? Ou bien allons-nous nous montrer enfin dignes de ces aïeux et dire calmement, mais fermement, aux nouveaux venus à quelles conditions ils peuvent entrer chez nous, à quelles conditions ils peuvent devenir Français et expulser sans faiblir tous ceux qui refusent de se plier à nos lois et à nos moeurs ? Puisque j'évoque devant vous nos aïeux, je voudrais finir en parlant du temps long, celui de l'histoire. Je vous le demande, mes chers collègues, dans quelle situation notre pays se trouvera-t-il dans dix, vingt ou cinquante ans si nous renonçons à affronter cette grave question migratoire qui se présente à nous ? Pensez-vous que ce sera toujours la France, de Louis XIV, de Napoléon ou de Charles de Gaulle ? La réponse, hélas, est dans la question ! Comme patriote français, comme parlementaire, j'ai honte de vous présenter aujourd'hui, mes chers collègues, un rapport sur une mission aussi manifestement mensongère.

d'asile (ADA), on ne comprend pas que le budget prévu pour 2020 soit de 444 millions d'euros, alors que la consommation pour l'année 2019 est à plus de 509 millions d'euros. Par quel hasard aurions-nous moins besoin d'attribuer l'ADA en 2020 qu'en 2019 ? Vous pariez sur le fait qu'il n'y aura pas de demandeurs d'asile supplémentaires en 2020.

vous faites le pari- nous voudrions être d'accord avec vous -qu'il faut augmenter les retours vers les pays d'origine, notamment en passant à 50 % et à 60 % des personnes placées en centre de rétention administrative.

le contexte de contrainte budgétaire, auquel nous sommes désormais malheureusement habitués, n'a pas empêché le Gouvernement d'augmenter, pour la troisième année consécutive, les crédits de la mission « Immigration, asile et intégration Ils s'établiront donc cette année à 1,8 milliard d'euros, en croissance de près de 130 millions d'euros, soit une augmentation de 8 % par rapport à la loi de finances initiale pour 2019. Ces moyens supplémentaires permettront d'atteindre les objectifs fixés par le Président de la République et le Premier ministre. Ils s'inscrivent dans le cadre des débats sur l'immigration qui se sont tenus le 7 octobre dernier à l'Assemblée nationale, puis le 9 octobre au Sénat dite « loi asile et immigration », laquelle est aujourd'hui pleinement entrée en application. Parallèlement, des mesures ont été annoncées par le Gouvernement le 6 novembre dernier dans le cadre du comité interministériel sur l'immigration et l'intégration. Pour tenir compte de l'accroissement des demandes d'asile, ce budget, qui vise la réduction des délais d'instruction à six mois des demandes d'asile de ressortissants de pays sûrs, prévoit une augmentation significative des effectifs de l'Ofpra et de la Cour nationale du droit d'asile. à renforcer également les capacités d'hébergement des demandeurs d'asile, car la constitution de campements insalubres de personnes migrantes dans le nord-est de Paris, que vous vous êtes engagé, monsieur le ministre, à évacuer d'ici à 2020, traduit aujourd'hui les dysfonctionnements de notre système d'hébergement et d'asile. Concernant la lutte contre l'immigration clandestine, s'il est vrai que les crédits qui y sont consacrés diminuent, cette baisse est à nuancer : nous le savons bien, ces crédits ne recouvrent pas la totalité des dépenses de l'État engagées dans ce domaine, lesquelles figurent également dans d'autres programmes. Enfin, permettre l'intégration des personnes que nous avons choisi d'accueillir dans notre pays est primordial. Cette hausse de 30 millions d'euros par rapport à l'année dernière permettra d'augmenter sensiblement le nombre d'heures d'enseignement de français et d'instruction civique, ainsi que les moyens dévolus à l'insertion professionnelle. Nous le savons tous, la maîtrise de la langue et l'emploi sont les fondements d'une intégration réussie. Je ne puis m'exprimer sur ce budget sans évoquer la situation dans mon département, qui, comme vous le savez, est fortement frappé par l'immigration illégale. La politique menée actuellement par le Gouvernement commence à produire des résultats encourageants, après des années d'incurie durant lesquelles les Mahorais étaient désespérés de constater que l'État avait pratiquement baissé les bras dans la lutte contre l'immigration clandestine. Le plan civilo-militaire de lutte contre l'immigration clandestine, dit « Shikandra », du nom d'un poisson qui mord quand on s'approche de son nid, traduit l'engagement pris par le Président de la République le 1 février 2019, lors du grand débat national à l'Élysée en présence des élus ultramarins. Lancée en août dernier par la ministre des outre-mer et par le ministre de l'intérieur, cette opération visait à atteindre les 25 000 reconduites à la frontière avant la fin de l'année 2019. Au 1 octobre, 22 000 reconduites avaient d'ores et déjà été réalisées. Conscient que cette immigration massive traduit un profond déséquilibre économique, le Gouvernement s'est également engagé à soutenir l'Union des Comores sur les questions de santé, d'éducation et d'agriculture en échange d'un réel effort dans la lutte contre les filières d'immigration et de traite d'êtres humains. Aussi, la première réunion du comité franco-comorien de haut niveau chargé d'assurer le suivi de la mise en oeuvre du document-cadre s'est tenue les 20 et 21 novembre dernier à Moroni. Récemment, dans un entretien du 13 novembre sur une chaîne de télévision française, le Président de l'Union des Comores a rejeté l'affirmation du Président de la République qui, en déplacement à Mayotte, rappelait que l'île était française. À cette même occasion, le Président comorien a déploré l'expulsion des immigrants illégaux depuis Mayotte vers les Comores. Il ne peut s'agir, à mon sens, que d'une posture, car le président Azali Assoumani sait bien que les termes de cet accord ne valent que si les engagements sont réciproques. Je dirai enfin quelques mots sur la situation migratoire de la Guyane, qui est également préoccupante. Elle a fait l'objet d'une récente mission de la commission des lois. Des expérimentations intéressantes sont en train d'être menées sur place, notamment sur le traitement de l'asile et sur la réorganisation de nos forces de sécurité.

Pour finir, ce budget nous semble allier fermeté et humanité. C'est la raison pour laquelle le groupe La République En Marche approuvera les crédits de cette mission. La parole est à Mme Esther Benbassa. Monsieur le Monsieur le président, monsieur le ministre, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, peu avant son élection à la présidence de la République, le candidat Macron louait la politique migratoire de Mme Merkel, qui avait « sauvé la dignité de l'Europe ». Par la suite, les accents humanistes utilisés sur la question de l'asile ont été remplacés par des gages à peine voilés aux populistes. Cela commence bien ! La première étape de cette évolution a bien évidemment été la loi « asile et immigration ». Depuis lors, les discours ambigus ont été multipliés et on parle désormais de quotas migratoires. La mission « Asile, immigration et intégration », telle qu'elle nous est présentée aujourd'hui, n'est d'ailleurs pas de nature à nous rassurer. En 2018, quelque 2 260 migrants sont morts noyés en Méditerranée. L'horreur que doit susciter ce chiffre devrait nous inciter à adopter des orientations financières diamétralement opposées aux PLF votés ces dernières années. Pourtant, le budget qui nous est soumis est particulièrement déséquilibré, tant la part belle y est faite au financement de la lutte contre l'immigration irrégulière, au détriment de l'intégration et de l'accès à la nationalité française. Le Gouvernement fait tout pour décourager les exilés de venir en France alors que ceux-ci fuient la guerre, la famine, les instabilités politiques et parfois même les dérèglements climatiques. Monsieur le ministre, une fois de plus- c'est le cas depuis 2015 -, vous minorez le nombre de migrants qui vont arriver sur notre territoire. De ce fait, les crédits de cette mission sont parfaitement sous-budgétisés. Vous revendiquez une politique migratoire dissuasive et inhumaine : ainsi, alors que près de 2 000 exilés sont sans logement dans la capitale, vous ne souhaitez pas créer de nouvelles places d'accueil en 2020. Dans le même temps, vous investissez 41,2 millions d'euros dans la création de centres de rétention administrative neufs, tout en refusant d'augmenter les budgets des prises en charge et d'accompagnement social des personnes retenues. Voilà qui en dit long sur votre volonté d'expulser et d'enfermer, plutôt que d'accueillir et d'intégrer. Finalement, la seule donnée positive de ce PLF est l'augmentation du budget de l'Ofpra, à hauteur de 20 millions d'euros. une disposition qui avait par ailleurs été demandée l'an passé par le groupe CRCE. M. Nunez nous avait alors opposé un refus catégorique. Ce budget est donc bien insuffisant ! Et il ne vient certainement pas rompre avec le désengagement de l'État, qui oblige les associations à compenser l'inaction des pouvoirs publics. Ainsi, je vous le demande, monsieur le ministre : à quand une politique migratoire digne, capable de répondre à cette crise de l'accueil ? À quand des places supplémentaires ouvertes aux primo-arrivants dans les centres d'accueil de demandeurs d'asile (CADA), afin de contrer la création de nouveaux camps de fortune dans nos rues ? À quand une aide juridique effective pour tous ces requérants, qui sont pris au dépourvu devant la complexité des procédures de l'Ofpra ? À quand une revalorisation de l'ADA et un meilleur accompagnement des migrants vers l'emploi ? Vous l'aurez compris, monsieur le ministre, nous ne cautionnons pas votre politique inique. En cohérence avec ses convictions, le groupe CRCE ne saurait voter ces crédits. Nous ne voulons ni de quotas de migrants économiques, ni de l'enfermement d'enfants dans les camps, ni de la répression des migrants aux frontières, ni de votre budget insincère ! La parole

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, « entre 2014 et 2019, les crédits affectés aux mesures d'éloignement des étrangers en situation irrégulière ont ainsi connu une progression limitée à 37,5

Je crois qu'il faut être vigilant et peut-être un peu plus nuancé. On pourrait croire que les crédits affectés aux mesures d'éloignement et le nombre de demandes d'asile sont liés alors qu'il s'agit pourtant de deux choses assez différentes. De ce fait, sur le sujet, la confusion quant aux notions de réfugiés, d'immigrés et d'étrangers est assez répandue. Il faut que nous prenions garde à ne à ne pas entretenir cette confusion- ce n'est pas si simple -et à ne pas faire le jeu des populistes. Pas de confusion, mais pas d'angélisme pour autant telle est la position du groupe Les Indépendants. Le sujet de l'immigration est une préoccupation majeure pour nos concitoyens, comme il l'est pour les Européens dans leur ensemble. Nous avons déjà eu l'occasion de rappeler que les réformes se sont succédé sur le sujet sans parvenir à apporter de solutions durables. Les migrations sont des phénomènes internationaux qui dépassent les seules sphères nationales. Il nous semble donc que c'est à l'Europe de se charger de la gestion des flux migratoires. Nous regrettons qu'elle n'ait pour le moment ni le mandat de remplir cette mission ni les moyens de le faire. L'espace Schengen est une chance pour tous les Européens. La liberté de circulation des individus, des marchandises et des capitaux a contribué à faire de notre continent un continent de paix et de prospérité. Cette liberté, qui fait notre force, ne doit pas se transformer en faiblesse. Il faut pour cela que l'Union se dote des moyens pour assurer le contrôle de ses frontières. L'augmentation du nombre d'agents Frontex y participe, mais elle est trop lente. Nous appelons aussi de nos voeux un changement de mentalités. L'Europe ne doit plus sous-traiter le contrôle de ses frontières. Nous avons vu que le refus d'assumer cette mission rend l'Europe vulnérable au chantage. Le comportement du président Erdogan en la matière est inacceptable. Nous ne pouvons tolérer d'être les otages de la Turquie, comme de tout autre pays. Le contrôle des frontières est une action qui nécessite parfois l'emploi de mesures coercitives. Quand certains seraient tentés de détourner le regard, il nous faut nous rappeler qu'il est nécessaire d'exercer cette mission et l'assumer. Il y va de notre souveraineté et de notre indépendance. La France doit prendre sa part, et nous saluons l'augmentation de plus de 7 % des crédits de la mission. Nous avons intérêt, tout comme les étrangers qui arrivent sur notre territoire, à ce que l'État consacre les moyens nécessaires au contrôle de l'immigration, pour que celui-ci se fasse dans les meilleures conditions. Les demandes d'asile, comme les deux rapporteurs l'ont rappelé, augmentent. Elles doivent être traitées dans les meilleurs délais, pour que les demandeurs qui ont vocation à en bénéficier puissent rester sous notre protection et que les autres quittent rapidement le territoire national. L'augmentation de 25 % des effectifs de l'Ofpra nous semble ainsi aller dans le bon sens. Nous regrettons en revanche la stagnation des crédits alloués à la lutte contre l'immigration irrégulière. Il nous semble en effet que c'est une priorité. Depuis trop longtemps maintenant, le taux d'exécution des obligations de quitter le territoire est inférieur à 25 %. Ce n'est pas acceptable. Quel message envoie-t-on en acceptant la violation de la très grande majorité des OQTF ? « Faire des lois Faire des lois et ne pas les exécuter, c'est autoriser ce que l'on veut interdire », disait Richelieu. Cela n'a pas changé ! En conclusion, nous ne souhaitons pas que la France se replie sur elle-même. Nous la voulons tournée vers le monde et vers l'échange. Mais nous souhaitons que cette ouverture soit encadrée par le strict respect de la loi. Il nous semble que c'est ainsi que nous pourrons faire face aux défis de l'immigration et de l'intégration : donnons-nous les moyens d'appliquer les lois.

souhaite être une force de proposition pour combattre le sentiment d'impuissance de l'État, qui est grave pour nos concitoyens, en matière de droit d'asile et de migration. Il s'agit de sujets qui touchent à l'essentiel, c'est-à-dire à la souveraineté

! Nous avons apprécié la volonté du Premier ministre il y a quelques semaines d'ouvrir un débat devant la représentation parlementaire sur ces questions.

renforcée », qui nécessite neuf pays. Nous sommes également très favorables à la renégociation de l'espace Schengen et à l'interopérabilité des systèmes d'information au sein des problèmes budgétaires. J'insiste sur ces questions numériques rien n'est réglé en cette matière, entre le système d'information Schengen (SIS), le système d'information sur les visas (VIS), le système entrée-sortie

En d'autres termes, si l'on veut vraiment avancer sur ce sujet, le meilleur service que l'on puisse rendre à notre pays ou à l'Europe est d'avoir une interface de recherche unique. Nous souhaitons également une simplification du droit de l'éloignement. Selon nous,

devant les juridictions administratives depuis trois ans- +38 000 requêtes -, dont 35 000 relèvent du droit des étrangers. Voilà très clairement

J'aurais mauvaise grâce d'oublier l'augmentation des moyens accordés à l'Ofpra. Ils sont considérables : +200 postes ! Je ne sais pas, mes chers collègues, si vous connaissez beaucoup d'agences ou d'autorités administratives indépendantes qui bénéficient d'un tel renforcement.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, l'asile est un droit, c'est aussi un devoir, car respecter le droit d'asile, c'est signifier ce que l'on souhaite comme société- une société qui respecte l'humanité, la liberté et la dignité de chaque personne. L'immigration, en revanche, est une politique, avec des principes, des objectifs et des moyens en cohérence. Malheureusement, de plus en plus, l'immigration est aussi le moyen de faire de la politique à partir des peurs, en les développant jusqu'à l'irrationnel. Dans ce jeu, certains sont actifs, développant la haine, stigmatisant les différences. D'autres sont passifs, craignant qu'une confrontation avec ce qu'ils pensent de l'opinion publique ne leur ferme la route du pouvoir.

N'ayons pas peur en parlant d'intégration. Mais, si l'on veut parler d'intégration, ne stigmatisons pas et ne confondons pas politique de lutte contre la fraude et politique d'intégration Pour être intégré, lorsque l'on est étranger dans un pays, il faut s'y sentir bien ; il ne faut pas se sentir différent. Je veux que mon pays réponde à cette exigence. Nous devons être attentifs aux droits des personnes en situation régulière,

aujourd'hui deux rendez-vous pour obtenir un récépissé provisoire à la suite d'une demande de renouvellement de titre de séjour. Ce document est obtenu quasiment au bout d'un an, c'est-à-dire au moment de son expiration.

peut entraîner. Il convient de veiller à ce que, dans le prochain cadre financier pluriannuel de l'Union européenne, les moyens de Frontex soient renforcés et que la participation française à cette agence soit importante

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, l'Europe connaît depuis 2015 une hausse significative des flux de migrants, obligeant les États membres à consentir des efforts financiers importants, à la fois pour traiter les demandes, accueillir les personnes dans des conditions convenables et lutter contre l'immigration irrégulière. La mission « Immigration, asile et intégration », dont nous examinons les crédits aujourd'hui, correspond en réalité à un peu plus de 20 % de l'ensemble des crédits alloués à la politique française de l'immigration et de l'intégration. Elle se décompose en deux programmes : le programme 303, « Immigration et asile », qui porte les crédits de garantie du droit d'asile et d'accueil des demandeurs d'asile ainsi que ceux qui sont liés à l'immigration irrégulière ; le programme 4, « Intégration et accès à la nationalité française », qui porte les crédits d'intégration des étrangers primo-arrivants et des réfugiés. On constate, à périmètre constant, une hausse de 9,8 % en crédits de paiement et de 6,3 % en autorisations d'engagement. Depuis 2017, il s'agit d'un quasi-doublement des crédits de cette mission. Tout d'abord, le projet de loi de finances prévoit des investissements significatifs pour faire face à la hausse de près de 22 % des demandes d'asile déposées en 2018. Les moyens de l'Ofpra

% du nombre d'équivalents temps plein. Ces efforts financiers permettront, je l'espère, de réduire le délai de traitement des demandes d'asile, qui est actuellement de plus de six mois. Je veux également saluer la hausse de plus de 7 % des crédits du programme 4, « Intégration et accès à la nationalité française », qui permet de financer la mise en oeuvre de l'intégration des étrangers en situation régulière, notamment le contrat d'intégration républicaine, le CIR, qui a été créé par la loi de 2016 et enrichi par la loi de 2018. Ce sont ainsi plus de 12 millions d'euros qui sont prévus dans ce projet de loi et qui financeront les formations linguistiques et l'insertion professionnelle. Néanmoins, je partage l'inquiétude de mes collègues de la commission des lois et de la commission des finances s'agissant des prévisions du Gouvernement en matière de demandes d'asile. Le scénario sur lequel est construit le projet de loi de finances repose sur la prévision d'une hausse de 12 % de la demande d'asile en 2019,

progresse de 33 % par rapport à 2019, elle reste inférieure aux crédits votés dans la loi de finances rectificatives de 2019 pour répondre, d'ores et déjà, aux besoins de cette année. Nul besoin d'être prophète pour savoir que l'enveloppe prévue dans le projet de loi de finances le sujet qui m'inquiète le plus reste l'hébergement des demandeurs d'asile. Actuellement, seul un demandeur sur deux est hébergé dans une structure appropriée. L'autre moitié est orientée vers l'hébergement d'urgence, destiné aux personnes en détresse, ou alors dans des hôtels qui ne répondent pas du tout à leurs besoins.

En effet, cette mission voit ses crédits diminuer de 26,39 % en autorisations d'engagement et de 9,98 % en crédits de paiement. Le Gouvernement explique cette diminution par la hausse significative des crédits alloués à cette politique dans le projet de loi de finances pour 2019, une augmentation qui avait pour objet de financer de nouvelles places de rétention, aujourd'hui en cours de construction, et dont les programmes sont en voie d'achèvement. Malgré cette hausse de 35 % des places en CRA depuis 2017, les chiffres restent alarmants : les taux d'occupation de ces centres sont en constante augmentation et atteignent en moyenne, pour le premier semestre 2019, un niveau d'environ 87 %. J'ai eu l'occasion de visiter le CRA de Vincennes il y a quelques mois et j'ai été bouleversée par les conditions de vie de ces femmes et de ces hommes, lesquelles ne sont pas conformes à l'idée que je me fais de la dignité humaine. C'est la raison pour laquelle je considère qu'une poursuite de l'effort amorcé l'an dernier aurait été plus que nécessaire. Enfin, je suis également surprise que les crédits alloués aux frais d'éloignement des migrants en situation irrégulière à l'issue d'une rétention stagnent à hauteur de 30 millions d'euros, alors que l'exécution réelle des décisions d'OQTF a atteint un taux historiquement bas de 15 %. Le groupe du RDSE souhaiterait que les débats se concentrent non pas sur des questions d'écritures comptables, mais sur les sujets de fond, et ils sont nombreux, ayant trait à la politique migratoire et d'asile qui est actuellement menée dans notre pays. Le budget présenté par le Gouvernement permettra-t-il de conduire la politique que celui-ci entend mener vis-à-vis des personnes étrangères présentes sur notre sol ? Sur le long terme, que dit l'évolution budgétaire du coût de cette politique ? Voilà deux questions qui nous préoccupent vivement. loi de finances que nous examinons prévoit en matière d'immigration, d'asile et d'intégration des efforts financiers timides et sûrement insuffisants. Cependant, ils ont le mérite d'exister.

car nous ne pouvons ignorer les préoccupations qu'elle suscite chez nos compatriotes. Bien sûr, elle interroge notre histoire, nos valeurs et notre modèle d'intégration, dans un contexte de crise économique et identitaire. Bien sûr, la France peut et doit s'honorer d'accueillir celles et ceux qui sont persécutés dans leur pays d'origine, mais avec dignité et dans le cadre d'un parcours d'intégration clairement défini. Bien sûr, cette question ô combien majeure ne date pas de 2017, et les réponses ne peuvent être franco-françaises ; il faut les envisager aussi dans le cadre européen, qui doit, d'ailleurs, être repensé.

Sur ce sujet, la réflexion relative à la réforme de l'aide médicale d'État (AME) a été lancée par le Premier ministre, et notre collègue Alain Joyandet en a proposé une traduction dans le cadre de ce projet de loi de finances. Si le Gouvernement tente de répondre au défi migratoire, il faut aller encore plus loin dans la lutte contre l'immigration illégale et le détournement massif du droit d'asile. La loi du 10 septembre 2018 pour à montrer ses effets, alors que les récentes propositions du Premier ministre conduiront nécessairement à la faire évoluer et ne répondent qu'à la partie émergée de l'iceberg. La hausse des crédits, pour la troisième année consécutive, dans le contexte budgétaire que nous connaissons va indéniablement dans le bon sens. Mais est-elle suffisante pour faire face à ces deux priorités ? Les 129 millions d'euros d'augmentation des crédits de la mission budgétaire seront, en réalité, absorbés en totalité par les 139 millions d'euros d'augmentation des crédits consacrés au droit d'asile. En outre, les crédits de paiement de la lutte contre l'immigration clandestine s'effondrent de 26,39 %, alors que c'est d'abord sur ce terrain qu'il nous faut porter nos efforts.

la pression migratoire, non pas seulement dans les préfectures, mais aussi dans nos collectivités, et le coût qu'elle représente au détriment d'autres politiques tout aussi indispensables et urgentes. À ce titre, le système de prise en charge des mineurs étrangers isolés ou non accompagnés est au bord de l'implosion, faute d'une politique publique à la hauteur. Depuis trop longtemps, l'État laisse les départements faire face seuls à une situation intenable toujours davantage de prise en charge et toujours moins de moyens. La réforme de la fiscalité locale, qui affaiblit les finances départementales, réduira encore davantage leurs marges de manoeuvre, déjà quasi La responsabilité juridique des présidents de départements sur ce sujet est d'autant plus inquiétante qu'ils sont obligés de la prendre en charge au détriment, parfois, d'autres enfants du département qui sont eux aussi en situation de détresse. Cela m'avait donné à l'époque de véritables sueurs froides, je puis vous l'assurer. Pour toutes ces raisons, la commission des lois du Sénat a donné un avis défavorable à l'adoption des crédits de la mission. Je partage l'analyse du président Philippe Bas sur la nécessité absolue de repenser notre politique d'immigration sur le fond. si notre pacte social implique que nous pouvons choisir qui accueillir sur notre sol, notre modèle républicain nous impose de le faire dans des conditions décentes, afin de garantir un parcours d'intégration réussi. Le nier, c'est faire le lit du communautarisme et du multiculturalisme, qui diluent la Nation. La parole Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues,

Les sénateurs présents ont gardé un souvenir poignant des frontières, des, envahis régulièrement par les migrants désireux d'aller en Angleterre. Il faut gérer efficacement cette misère humaine et lutter contre les trafics d'êtres humains.

constat d'évidence que les sujets ayant trait à l'immigration devaient être traités par les différents États européens. Chaque pays est concerné par l'exaspération de sa population. Les citoyens français restent très touchés par les problèmes humains que connaissent les populations migrantes. Pourtant, en même temps, leur exaspération s'amplifie, en raison de l'indécision des gouvernements jamais su concilier humanité et fermeté dans l'application de la loi. La lutte contre la traite des êtres humains ne semble pas être efficace. La lutte contre l'immigration irrégulière, disons-le, est un échec.

soit parce que l'OQTF est annulée par le juge administratif pour vice de forme, soit parce que l'administration n'a pas été en mesure d'organiser son éloignement dans les délais impartis. Le coût humain et financier de cette politique n'est pas acceptable. Nous avons ainsi accompagné la commission d'enquête sur l'état des forces de sécurité intérieure à Lesquin, dans le Nord, où le centre de rétention administrative gère les individus en attente de connaître leur sort. Il est particulièrement choquant que des personnes en situation irrégulière se maintiennent sur le territoire. Pourtant, la crédibilité du pouvoir exécutif

En contrepartie des moyens qu'on se donne en matière d'intégration, il faut être très ferme avec les personnes en situation irrégulière. Sinon, il n'y a aucune raison pour que celles en situation régulière fassent des efforts pour s'intégrer.

Jamais il n'a été aussi haut, puisqu'il a progressé de 18 % cette année. Votre remarque sur les relaxes systématiques de passeurs est assez éloignée de la réalité, et j'en ai été surpris. Je

Les crédits de la mission « Immigration, asile et intégration » sont en cohérence avec nos ambitions. C'est pourquoi ils s'établiront, en 2020, à 1,82 milliard d'euros, soit une augmentation de 9,6 % à périmètre constant.

Parmi elles, 90 000 sont arrivées par la voie du regroupement familial ; ce chiffre est stable depuis de très longues années. Nous notons l'arrivée de 83 000 étudiants et de 33 000 personnes pour des motifs économiques. Ces deux dernières catégories sont en augmentation.

améliorer la rapidité de la décision que nous devons à celles et ceux qui font une demande de protection. Il n'est pas normal qu'un Géorgien venu

Nous avons fait des efforts sur ce point, et devons les poursuivre. L'immigration, l'asile et l'intégration ont été au coeur de l'action du Gouvernement depuis la première minute du quinquennat, mais avec lucidité et sans angélisme. Nous menons une politique claire, ferme, ambitieuse.

à venir, l'exécutif justifie la sous-budgétisation et l'insincérité des moyens de la mission « Immigration, asile et intégration » par une prévision erronée de stagnation du nombre de demandeurs d'asile en 2020. Mes chers collègues, je sais que vous êtes d'accord avec moi sur cette question, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle la commission des lois a refusé de voter les crédits de ce budget. La crise de l'accueil, que nous connaissons, n'est pas près de s'arrêter. Les flux migratoires vont se poursuivre, et nous ne sommes absolument pas prêts à les recevoir.

et des professionnels du droit des migrants. Nous ne pouvons pas accepter l'installation de nouveaux camps de fortune dans nos rues. Les bidonvilles qui ont proliféré à Calais ou aux portes de la Chapelle et d'Aubervilliers sont des hontes humanitaires pour notre pays. En refusant d'accorder davantage de moyens aux centres d'hébergement, le Gouvernement se fait complice de la souffrance des 2 000 exilés sans domicile qui errent dans les rues de la capitale. Afin de corriger cette carence, le présent amendement vise à consacrer 20 millions d'euros à la création de 2 000 nouvelles places dans les centres d'hébergement d'urgence. Quel

l'ensemble des fausses informations qui circulent sur notre capacité à intégrer et à accepter toute la misère du monde. Qui parle aujourd'hui du contournement du droit d'asile ? C'est le Président de

de ces personnes, qui ont accompagné nos efforts en Afghanistan.

réfugiés (Diair). Normalement, les logements sont fournis par l'armée et l'accompagnement social réalisé par des opérateurs financés par notre ministère. Nous portons donc une attention toute particulière, et bien légitime, sur cette situation, tant il est nécessaire que nous soyons en cette affaire à la hauteur de notre propre histoire.

J'apprécierais que les prochains avis de la commission soient étayés par des chiffres, des arguments juridiques, des discussions sur la réalité et non sur des jugements de valeur arbitraires.

Il est un fait que la France est devenue le premier pays pour les demandes d'asile. C'est bien le signe qu'elle est le maillon faible

en réalité, que c'est toute la politique migratoire qu'il faut remettre sur la table. Comment faire pour mieux intégrer ceux qui sont en France de manière régulière, ceux qui obtiennent le statut de réfugié, en mettant vraiment les moyens sur l'intégration. Et comment faire pour que ceux qui n'ont pas à être sur le territoire national n'y soient pas ?

Karoutchi. Vous avez raison, monsieur le ministre, quand vous êtes un véritable demandeur d'asile, que vous avez été persécuté chez vous, que, pour venir en Europe, vous avez

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je voudrais revenir sur les faits, parce

madame Goulet,

l'an passé. Cela étant, ce qui était valable hier n'est plus suffisant aujourd'hui. Dans un contexte marqué par une demande d'asile soutenue et par une immigration en progression, les moyens budgétaires prévus par l'exécutif pour 2020 sont tout simplement insuffisants. Partant de prévisions erronées concernant le nombre de demandes d'asile que devra traiter l'Ofpra, l'exécutif a déterminé le montant des crédits en retenant l'hypothèse d'une stabilisation de la demande d'asile en 2020. Ce calcul inexact entraîne un risque de sous-budgétisation de la mission et, oserais-je dire, une insincérité budgétaire. Cette hypothèse est jugée irréaliste par l'ensemble des associations et organismes compétents, estimant que l'Ofpra risque l'engorgement, du fait d'un nombre croissant de requérants dans les années à venir. Ainsi, nous jugeons nécessaire d'accroître encore davantage le budget de cet Office, à hauteur de 5 millions d'euros. Cette augmentation a pour objectif d'assurer la formation et le recrutement de plus de personnel qualifié

selon l'ONU, le nombre de personnes migrantes qui se sont noyées en mer en 2018. Ainsi, année après année, la Méditerranée se transforme en cimetière. Les exilés sont arrachés à leur terre natale par les affres de la vie, par les guerres ou par les instabilités politiques et ils n'aspirent qu'à une chose : trouver la paix en Europe, en attendant de pouvoir retrouver leur pays d'origine, une fois que l'Afrique et le Moyen-Orient auront été pacifiés. Du fait de notre inaction coupable, nombre d'entre eux n'atteignent jamais les côtes européennes. Il est temps que cela cesse, que nous portions assistance à ces femmes et à ces enfants naufragés,

venu remplacer l', pour venir en aide aux exilés se trouvant en détresse en Méditerranée. Tel est l'objet du présent amendement : demander l'octroi de 5 millions d'euros à cet effet. Les mécanismes européens d'aide aux naufragés ne sont pas suffisamment effectifs et la France se doit d'être à la la pointe de la solidarité à l'endroit des migrants. Quel

du Gouvernement ? Madame la sénatrice, la France est au rendez-vous de la solidarité. Depuis que je suis aux responsabilités au ministère de l'intérieur, notre pays est le premier pays européen en capacité et en offre d'accueil

Je vous soumets la problématique globale : on dénombre actuellement 660 000 réfugiés ou demandeurs du statut de réfugié en Libye, on pourrait donc considérer qu'il serait logique d'accueillir ces 660 000 personnes en France. Ce n'est pas la position de la France.

avec le plus grand cynisme, des personnes qui sont dans le malheur et qui, parfois, ont rassemblé toutes les économies du village pour payer le prix permettant de tenter d'arriver en Europe.

devons faire en sorte que ces trafics cessent et que les trafiquants soient sanctionnés comme ils le méritent ; ce sont des gens qui, de manière cynique, je le répète, jouent avec la vie des êtres humains.

Plusieurs associations et plusieurs praticiens du droit des migrants que nous avons entendus ont porté à notre attention de nombreux cas de migrants atteints de troubles psychotraumatiques. L'indifférence du Gouvernement sur ce grave enjeu de santé publique nous déconcerte. La souffrance psychique des migrants est directement provoquée par les violences que subissent ces personnes, tant dans leurs pays d'origine que lors de leur traversée vers l'Europe. Ces multiples troubles, parmi lesquels figure le syndrome de stress post-traumatique, compliquent également le travail des agents de l'Ofpra, censés examiner la véracité des récits et témoignages. Les demandeurs d'asile qui en sont atteints souffrent d'amnésie traumatique et ne peuvent relater aisément et avec précision les persécutions subies. Ces pathologies mentales peuvent être plus graves encore. Sans suivi médical, les individus peuvent pâtir à long terme de maladies psychiatriques de plus grande ampleur, comme la schizophrénie. Parce que le suivi psychotraumatique est inexistant et occulté par les politiques publiques, nous proposons la création d'un fonds doté de 1 million d'euros, destiné à la prise en charge des pathologies dont souffrent ces personnes brisées par l'exil. Mes chers collègues, il est de notre devoir de mettre en place, au sein de notre politique d'accueil et d'intégration, une offre plus ample de soins en santé mentale, afin de redonner confiance et dignité à ceux qui sont atteints de syndromes psychotraumatiques.

Monsieur le ministre,

Monsieur le ministre,

Cela aboutirait à priver 6 000 personnes des cours d'apprentissage du français. Il me semble malvenu de ne pas faire bénéficier ces personnes des moyens d'intégrer la République. Ce dernier article rattaché à la mission est un bel exemple de ce que nous subissons en France, sur l'ensemble du territoire.

ministre. Le ministère de l'intérieur va être chargé de gérer les mutualisations des fonctions support des services déconcentrés de l'État. Il a tiré son épingle du jeu dans un processus de réorganisation des services déconcentrés inauguré par son refus de délaisser ses emplois et ses moyens au profit du Premier ministre. On peut donc dire que « la force a fait l'union » ! Jacques Genest, que je remplace aujourd'hui, s'étonne avec moi que les crédits de fonctionnement et d'investissement n'aient pas encore suivi les emplois. Nous relevons que certaines administrations essentielles restent à l'écart des réorganisations en cours.

Oui ! ... la commission des finances est sensible aux perspectives ouvertes par les restructurations des états-majors régionaux, mais déterminée à obvier à toute nouvelle paupérisation de l'État de proximité.

Ce programme résulte de la fusion de l'ancien programme 307, « Administration territoriale », qui rassemblait les moyens des préfectures, des sous-préfectures et des représentations de l'État dans les territoires d'outre-mer, et du programme 333, Moyens mutualisés des administrations déconcentrées », qui regroupait les crédits des divers ministères supportant notamment les directions départementales interministérielles, les délégations régionales placées sous l'autorité des préfets de région et les secrétariats généraux pour les affaires régionales. Grâce à ce jeu de bonneteau budgétaire, qui frise, en cette occasion, la perfection, les moyens consacrés à l'administration territoriale apparaîtront en forte hausse à un lecteur un peu rapide, avec 2 460 millions d'euros d'autorisations d'engagement, soit une augmentation

Ces augmentations en trompe-l'oeil sont l'effet du transfert de moyens existants, jusque-là comptabilisés hors du périmètre du ministère de l'intérieur, au titre des missions interministérielles. Ce petit jeu annuel de brouillage des « périmètres » des missions et des programmes, pour le dire dans le patois des bureaux, ne permet plus au parlementaire ordinaire de suivre les redistributions de crédits.

Loin de marquer une rupture, le projet de loi de finances pour 2020 poursuit la politique constante de dissolution de l'administration territoriale de l'État.

Jérôme Bascher, cela est notamment dû au changement de périmètre de la mission. Le programme 333, « Moyens mutualisés des administrations déconcentrées », fusionne avec le programme 307, « Administration territoriale », ce qui élargit la mission dans son ensemble et augmente ses crédits.

Tout d'abord, je tiens à saluer l'intéressante mutualisation des moyens opérée sur plusieurs programmes. Elle doit se traduire par une amélioration de la qualité des services. J'en profite pour répéter que des services de proximité dont l'accessibilité est facilitée et la qualité renforcée

Alors que cette réforme se poursuit, la phase de réduction d'emplois prévue pour les missions non prioritaires est achevée ; elle a été très importante. L'étape de redéploiement des emplois en direction des missions prioritaires n'est, elle, pas terminée. Les ajustements sont en cours. Je souhaite que ces évolutions soient guidées par un souci d'amélioration de la qualité des services. Je répète que l'institution préfectorale est indispensable à notre pays et aux services rendus à nos concitoyens. La baisse de ses effectifs ne doit pas entraver son action ni accentuer le sentiment d'éloignement de certains territoires très ruraux. L'année dernière, j'ai souligné le rôle du préfet de Maine-et-Loire et son action particulière dans le cadre d'une prise d'otages. Le PPNG a également permis de remodeler la délivrance des titres tels que les passeports, les cartes nationales d'identité ou encore les permis de conduire. Ce réaménagement a été fortement orienté sur la dématérialisation. Sur ce point, l'entrée du numérique dans les procédures est une bonne nouvelle. Cependant, elle n'est pas tout le temps efficace ; surtout, certains territoires ruraux s'en trouvent défavorisés. Nous devons donc faire attention à ne pas accentuer les fractures entre nos territoires. Enfin, je souhaite porter la lumière sur un dernier point de ce programme, qui me semble particulièrement important : la baisse du budget du contrôle de légalité et, surtout, du conseil aux collectivités territoriales. Cette activité

Concernant les autres programmes, le budget du programme 232, « Vie politique, cultuelle et associative », prévoit une enveloppe de 132 millions d'euros réservée aux élections municipales. Les montants alloués au soutien aux formations politiques restent les mêmes, ce qui est récurrent. Quant au programme 216, « Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur », il bénéficie de l'augmentation importante des crédits alloués à la mission, notamment en raison de la création de nouvelles directions et agence. Un budget cohérent et raisonnable est positif à la fois pour l'État et pour les collectivités territoriales, surtout lorsque son périmètre s'élargit. La place centrale du corps préfectoral doit être accompagnée de moyens suffisants

et encore plus sur les maisons France Services annoncées par le Gouvernement. Au reste, cette annonce n'a rien d'extraordinaire, puisque c'est la suite d'un processus déjà engagé. Cependant, monsieur le ministre, je veux, une fois de plus, appeler votre attention sur la réalité des territoires ruraux

sont victimes d'une double peine résultant de la dématérialisation rapide et systématique de nombreuses procédures et des formalités administratives ainsi que de l'absence de mobilité

de l'état civil (Comedec). Lors de son audition, le 26 juin dernier, Jean Michel Brevet, chef de la division de l'expertise en fraude documentaire, relevait les failles de ce système Un autre problème particulièrement répandu en France est aussi la détention frauduleuse d'un document authentique sur la base de faux justificatifs. C'est un point faible à la fois pour les titres de séjour et à la fois pour les documents français. Pour les titres de séjour, on n'a jamais voulu imposer

Monsieur le président, monsieur le ministre, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, au travers de la mission « Administration générale et territoriale de l'État », le ministère de l'intérieur met en oeuvre trois de ses responsabilités fondamentales : : garantir l'exercice des droits des citoyens, assurer la présence et la continuité de l'État sur le territoire, mettre en oeuvre à l'échelon local les politiques publiques nationales. De fait, cette mission interroge les moyens que se donne l'État pour répondre à un double enjeu : celui de la démocratie et celui de la proximité. S'agissant des moyens, la mission change d'échelle,

L'administration territoriale de l'État est désormais concernée par le cadre du programme de réformes « Action publique 2022 », qui vise à dessiner une nouvelle organisation déconcentrée. S'il est prévu un mouvement de balancier vers les départements, des efforts budgétaires importants sont demandés aux administrations déconcentrées. Certes, l'État doit se recentrer et en finir avec un réflexe « touche-à-tout », dont il n'a plus les moyens- nous sommes tous d'accord sur

des procédures est indispensable. Toutefois, le baromètre du numérique indique qu'un Français sur trois n'a pas eu recours à l'e-administration en 2017. Pour sa part, France Stratégie évalue à 14 millions le nombre de Français éloignés du numérique. C'est bien parce qu'il est nécessaire de prendre en compte la fracture numérique et « l'illectronisme », au regard du principe républicain d'égalité devant le service public, que la stratégie nationale pour un numérique inclusif a été actée

Là encore, l'avenir nous dira ce qu'il en est. La mission aborde également la question du rapport entre l'État et les collectivités locales. Il ressort que des efforts budgétaires sont demandés, notamment sur le contrôle de légalité et le conseil aux collectivités. Malgré le resserrement des actes à transmettre au contrôle de légalité, les conséquences de l'extension du rescrit administratif aux collectivités prévue dans le projet de loi Engagement et proximité ? De même, l'affectation de 30 équivalents temps plein à la future Agence nationale de la cohésion des territoires nous laisse quelque peu songeurs.

Cette fusion permet au Gouvernement de présenter une hausse en trompe-l'oeil du programme, dénommé à présent « Administration territoriale de l'État ». En effet, comme vous l'aurez compris, mes chers collègues, la hausse résulte, en réalité, de transferts de crédits. Ce que l'on peut dire, c'est que le budget de la mission « Administration générale et territoriale de l'État » reste le parent pauvre du Mis à part le changement de périmètre, dont je viens de faire état et qui a entraîné une hausse mécanique des crédits, le budget de la mission reste globalement stable, avec une hausse de 50 millions d'euros, en grande partie due aux élections municipales du mois de mars prochain et à la création de la nouvelle direction du numérique. Pourtant, dans nos territoires, ce à quoi nous assistons, c'est à un recul des services publics, surtout des services de proximité. La dématérialisation à marche forcée a conduit à la suppression de nombreux points de contact qui permettaient à une population souvent âgée

de services au public pour 2 054 cantons. Ce sont donc plus de 700 maisons France Services qui doivent être déployées. Or aucun financement n'est prévu dans le projet de loi de finances, car le Gouvernement mise sur des mutualisations avec des structures préexistantes. En fin de compte, je crains fort que ce projet ne soit mis à la charge des collectivités territoriales, qui financent déjà la moitié des actuelles MSAP. Dans la même veine, à la suite du plan Préfectures nouvelle génération, qui a dématérialisé les demandes de délivrance de titres et qui a connu des dysfonctionnements majeurs, le Gouvernement annonce, pour 2020, la création de secrétariats généraux communs aux services préfectoraux et aux services déconcentrés, création qui justifie la fusion des programmes que j'ai déjà évoquée. Je tiens à rappeler que, si cette dématérialisation est certainement nécessaire au vu des évolutions technologiques, elle ne doit pas accroître la fracture numérique territoriale et sociale. Le Défenseur des droits a d'ailleurs, dans son rapport de l'année dernière, proposé de ménager des voies alternatives non dématérialisées pour faciliter l'accès du droit à tous.

devait y remédier, en offrant un guichet unique et des moyens opérationnels pour les porteurs de projets dans les territoires. Or on ne peut que noter la faiblesse des moyens financiers dédiés à cette agence dans le projet de loi de finances pour 2020, avec un budget de 50 millions d'euros, soit trois fois moins que le

L'agence ne pourra pas, sans nouvelles recrues, travailler mieux que ne le font actuellement les structures préexistantes, qui souffrent- c'est notamment vrai pour le CGET -d'une réputation défavorable. Il y aura donc encore une fois moins de personnes pour travailler en faveur des territoires ruraux et fragiles Un autre sujet préoccupe les élus locaux que nous sommes : les effectifs du contrôle de légalité et du conseil, qui accusent une baisse de 174 ETP sans qu'aucune explication soit fournie. Les moyens budgétés sont diminués de 21 %, alors que les municipalités ont de moins en moins de moyens financiers pour traiter les problèmes juridiques, qui sont pourtant, eux, de plus en plus nombreux.

ne nous satisfait pas, dès lors que le phénomène sectaire va bien au-delà du seul phénomène religieux et concerne également le monde associatif, professionnel, médical, culturel et sportif. Cette décision est d'autant plus incompréhensible que la Cour des comptes avait pourtant signalé que les ressources de la Miviludes, au demeurant très modestes puisqu'elles sont de moins de 500 000 euros, avaient été sensiblement réduites au cours des dix dernières années. Mes chers collègues, les sénateurs de mon groupe et moi-même ne nions pas la nécessité de réduire la dépense publique afin de ne pas mettre en péril notre économie. Néanmoins, nous déplorons que ce soient toujours les mêmes secteurs qui en pâtissent. Nous déplorons ainsi le recul sans accompagnement et sans explication de l'administration dans nos territoires. Ce projet de loi de finances n'accorde de moyens supplémentaires ni à nos préfectures et sous-préfectures ni aux administrations déconcentrées qui ont été rattachées à cette mission.

programme 354, « Administration territoriale de l'État » découle de la fusion, au 1 janvier, du programme 307, « Administration territoriale », et du programme 333. Le premier recouvrait l'ensemble des moyens des préfectures, des sous-préfectures et des représentations de l'État dans les collectivités d'outre-mer ; le second regroupait les crédits de fonctionnement des directions départementales interministérielles, des directions et délégations régionales placées sous l'autorité des préfets de région et des secrétariats généraux pour les affaires régionales, et portait également les emplois déconcentrés gérés par les services du Premier ministre. Cette fusion au sein au sein d'un même programme nous fait perdre un peu de visibilité cette année. Nul doute qu'elle traduit une volonté de cohérence et d'efficacité et qu'elle nous donne la lisibilité exigée constitutionnellement pour l'avenir. du programme 354 s'accompagne de deux évolutions majeures : l'extension du périmètre de l'ancien programme 333 à l'outre-mer et la prise en charge de l'ensemble des emplois issus des préfectures et des directions départementales interministérielles, qui seront affectés aux secrétariats généraux communs. Là encore, cohérence et efficacité. efficacité. Il est ardu de comparer les crédits de ce programme avec 2019, le périmètre n'étant plus le même. Toutefois, ce programme a été l'objet ces dernières années de réformes importantes.

sont d'abord par la mise en place de circuits de gestion efficaces permettant de renforcer leur dimension déconcentrée, participant ainsi à la mise en oeuvre de la réforme de l'organisation territoriale. Elles le sont ensuite par l'accompagnement à la création des secrétariats généraux communs. Ces structures interministérielles devront être créées dans chaque département avant le 30 juin 2020. Elles amélioreront la qualité des services rendus. Les Les priorités sont enfin renforcées par la poursuite du plan Préfectures nouvelle génération, qui consiste à repenser les modalités de délivrance des titres aux usagers en s'appuyant sur la dématérialisation des procédures. Là encore, cohérence et efficacité.

Le programme comprend également le financement de la vie politique à travers l'attribution de l'aide publique aux partis et au remboursement des frais de campagne des candidats. En matière de vie associative et cultuelle,

Enfin, les dépenses du plan de lutte anti-terroriste supportée par le programme 232 permettront l'ouverture de nouveaux diplômes universitaires et le financement de programmes de recherches académiques sur l'islam.

Cette nouvelle direction a pour vocation de répondre aux objectifs de transformation numérique dans l'ensemble des politiques publiques assumées par le ministère de l'intérieur et de proposer ainsi plus d'efficacité et de services aux usagers. J'en viens aux services aux usagers. Dans son rapport, notre collègue Jacques Genest semblait dubitatif quant à l'effectivité de l'annonce faite par le Président de la République concernant les maisons France Services : il craignait qu'elles ne se transmuent en coquilles vides.

En outre, la Banque des territoires de la Caisse des dépôts et consignations investira, d'ici à 2022, 30 millions d'euros pour assurer le déploiement des maisons France Services, avec notamment deux objectifs

Le groupe CRCE, qui a toujours milité pour un renforcement des moyens d'une fonction publique territoriale en capacité d'assurer la présence physique de la République dans l'ensemble du territoire- y compris à Forcalquier - ne peut que soutenir la position de la commission des lois. Il le fait d'autant plus volontiers que ce désengagement continu de l'État vis-à-vis des territoires est particulièrement évident en matière d'ingénierie publique,

ce qui n'empêche pas le Gouvernement d'afficher régulièrement son intention de répondre aux attentes fortes des petites collectivités. Le nouveau report de la cartographie de l'offre d'ingénierie publique et privée, demandée au préfet au mois de mars 2016, est bien le signe que le Gouvernement n'a aucune intention d'honorer ses engagements. Ces retards et ces tergiversations auraient pour origine, nous dit-on, la mise en place, toujours attendue, de l'Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT), dotée- ai-je cru comprendre -de pseudopodes locaux, pilotés, comme on l'imagine faute de précisions officielles, par les préfets. D'où une première interrogation : de quelle ingénierie parle-t-on ? De l'accompagnement des collectivités dans la définition de leurs projets territoriaux,

Autant de bonnes raisons pour le groupe CRCE de ne pas voter les propositions budgétaires relatives à la mission, la principale étant que la fonction publique territoriale est absolument indispensable à la présence de la République sur le territoire. C'est une

elle a une incidence directe et très concrète pour nos compatriotes dans nos territoires, surtout les plus ruraux d'entre eux. Elle porte en effet sur les crédits nécessaires au fonctionnement des préfectures, au pilotage des politiques du ministère de l'intérieur et à l'exercice de la citoyenneté : élections, vie politique et culte. La hausse de près de 18 % des crédits qui sont affectés à cette mission, prévue par le projet de loi de finances pour 2020, tient principalement à deux réformes : d'une part, la création d'une direction du numérique et la poursuite d'investissements en matière de systèmes d'information et de communication ; d'autre part, la mise en place, au cours de l'année 2020, des secrétariats généraux communs aux préfectures et aux directions déconcentrées interministérielles. Cette dernière réforme s'inscrit dans la poursuite des objectifs fixés par le programme Action publique 2022. Ainsi, en réalité, au-delà des transferts purement comptables, cette mission voit son budget stabilisé à 4 milliards d'euros. Cela appelle trois observations principales. La première observation a trait à la présence de l'État dans nos territoires. En effet, si le processus, sans doute souhaitable, de mutualisation et de dématérialisation se renforce, face à des citoyens qui demandent à l'administration des réponses claires et adaptées à leur situation personnelle, il ne peut se faire dans le même temps toute sa place à l'État pour assurer le respect des principes républicains d'égalité devant le service public dans l'ensemble du territoire national. L'État doit entendre le sentiment d'abandon de nombreux habitants des territoires ruraux, alimenté par les suppressions successives des relais physiques de l'État dans leur commune au profit des services en ligne ou éloignés des bassins de vie.

pour anticiper le désengagement de l'État lors du quinquennat précédent en préservant leur présence territoriale. La deuxième observation concerne le dynamisme de la démocratie locale. En effet, le programme 232, « Vie politique, cultuelle et associative », inscrit dans cette mission, assure l'exercice de la démocratie par le biais des crédits notamment dédiés à l'organisation des élections. Chacun a en mémoire, surtout dans cette assemblée, le renouvellement des conseils municipaux au mois de mars prochain. Or, comme ancien maire, je sais à quel point le projet de loi Engagement et proximité suscite des attentes fortes, tant les défis des élus locaux sont proportionnels à leur courage et à leur engagement au service de leurs administrés. La crise des vocations, la complexité administrative,

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le champ de la mission « Administration générale et territoriale de l'État » est très large. Selon les termes du projet annuel de performance (PAP), au travers de cette mission, le ministère de l'intérieur met en oeuvre trois de ses responsabilités fondamentales garantir l'exercice des droits des citoyens dans le domaine des grandes libertés publiques, assurer la présence et la continuité de l'État sur l'ensemble du territoire de la République, mettre en oeuvre à l'échelon local les politiques publiques nationales. De manière plus pragmatique, la mission porte sur la délivrance des titres sécurisés, le contrôle de légalité, l'accueil des migrants, le plan Préfectures nouvelle génération, etc. La liste étant très longue, je m'arrêterai seulement sur trois sujets. de finances pour 2020 portent la création d'une direction du numérique qui rassemblera différentes directions réparties dans les services du ministère de l'intérieur, voire relevant d'autres ministères. Pas moins de sept programmes budgétaires sont concernés par cette création. Rattachée au secrétaire général, cette structure aura pour mission de piloter les projets informatiques transversaux, les réseaux de télécommunications professionnels, les applications relatives aux élections ainsi que le répertoire des associations. Cette nouvelle direction, monsieur le ministre, pourrait utilement se saisir du problème de la transmission des procurations entre les commissariats, les tribunaux d'instance et les communes. Comme M. Jérôme

Genest, porte un avis circonspect sur cette agence : « Avec l'Agence nationale de la cohésion des territoires, on crée une énième agence. Nous verrons bien le service que ça rendra à la population et aux collectivités territoriales. Je me souviens avec une certaine nostalgie de l'élan donné à l'aménagement du territoire par la Encore une fois, nous verrons ce qu'il en sera, et si les 30 équivalents temps plein travaillé (ETPT) prévus apportent un plus. » Avant même son entrée en service, il me semble que cette agence souffre d'une incohérence : toutes les associations représentatives des collectivités auront un représentant au sein du conseil d'administration, toutes

Enfin, j'en viens au projet de maisons France Services. Comme le souligne avec justesse le rapporteur spécial, nous avons les annonces et nous n'avons pas les financements. En effet, si j'en crois le site www.gouvernement.fr, l'objectif est de labelliser un maximum de maisons France Services d'ici à la fin de cette année, en visant en priorité les zones rurales et les quartiers prioritaires de la ville. L'objectif fixé par le Premier ministre est que 300 maisons France Services soient pleinement opérationnelles d'ici à 2020 et une par canton L'État et ses partenaires contribueront au fonctionnement de chaque maison à hauteur de 30 000 euros par an. Or le PAP de la mission ne fait nullement mention des maisons France Services. Ce constat factuel laisse circonspect sur les moyens financiers mis au service de cette ambition. Pour toutes ces raisons, le groupe Les Républicains se rangera à la sagesse du Sénat.

parole est à M. le ministre. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, l'examen des crédits de la mission « Administration générale et territoriale de l'État » est toujours une étape importante.

Ce budget est donc une partie de la réponse du Gouvernement à cette soif de justice territoriale exprimée voilà un an. Je le dis fermement : les territoires abandonnés par la République, cela n'existe pas.

Les réformes engagées cette année, notamment celle de l'administration territoriale de l'État, démontrent la confiance qui a été placée dans le ministère de l'intérieur pour assurer cette présence. Ainsi est renforcée la place des préfets de département dans le pilotage et dans la coordination des politiques publiques de l'État dans les territoires.

1,8 milliard d'euros sont ainsi consacrés à l'administration territoriale de l'État et 1,41 milliard d'euros à l'administration centrale. Au-delà de ces chiffres, l'année 2020 verra l'aboutissement de plusieurs réformes majeures pour le ministère de l'intérieur,

l'État se réorganise en profondeur et que des services qui dépendent des services du Premier ministre sont confiés au ministère de l'intérieur, cela crée inévitablement des mouvements budgétaires. Nous ne les avons pas cachés : nous les avons présentés au contraire en détail dans les documents budgétaires qui vous ont été remis.

des préfets, le ministère de l'intérieur sera ainsi en mesure de mieux piloter la présence de l'État dans les territoires. Ce nouveau programme accompagne une réforme importante localement : je veux parler de la création des secrétariats généraux communs pour les services de l'État dans les préfectures.

monsieur le ministre,

L'exercice effectif de ce nouveau droit constitutionnel par les citoyens implique que ceux-ci soient dûment informés de son existence et de ses modalités. Or le Gouvernement a décidé de s'en tenir à la stricte obligation de la mise en oeuvre de la plateforme de recueil des signatures prévue par les textes.

par lui-même, que des mesures soient nécessairement prises, notamment par le Gouvernement, pour assurer l'information des électeurs sur l'existence » d'un référendum d'initiative partagée. Je suis d'autant plus libre de le dire, madame Harribey, que,

qui est magnifiée par la réponse de M. le ministre de l'intérieur, lequel ne manque pas de se référer à des épisodes historiques que j'ai quelques raisons de bien connaître. On peut penser ce que l'on veut de l'article 11 de la Constitution. Je pense d'ailleurs qu'il serait urgent de le réformer, ce qui supposerait, monsieur le ministre, qu'une révision constitutionnelle soit cas, l'article 11 existe et, si l'on parle non pas d'hier ou d'avant-hier, mais d'aujourd'hui, chacun peut voir qu'il y a deux poids, deux mesures